La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 2 mai 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? Monsieur le président, lors du scrutin n° 87, portant sur l'ensemble de la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, M. Alain Bertrand a été enregistré comme s'étant abstenu, alors qu'il souhaitait voter pour.

Mes chers collègues, par lettre en date du lundi 6 mai 2019, le Gouvernement sollicite l'inscription à l'ordre du jour du Sénat du lundi 27 mai, après-midi et soir, et, éventuellement, du mardi 28 mai, après-midi et soir, du projet de loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet. Nous pourrions entamer l'examen de ce texte en séance publique le lundi 27 mai, à seize heures. La réunion de la commission pour établir le rapport et le texte est fixée au mercredi 22 mai, au matin. Le délai limite pour le dépôt des amendements de séance pourrait, quant à lui, être fixé au vendredi 24 mai, à midi. Y a-t-il des oppositions ? ... Il en est ainsi décidé. Par ailleurs, à la suite de la nomination de M. François Pillet au Conseil constitutionnel et de la démission de Mme Catherine Troendlé de son poste de juge suppléante, le scrutin pour l'élection d'un juge titulaire et d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République pourrait se tenir mardi 14 mai, de quatorze heures trente à quinze heures, en salle des conférences. Le délai limite pour le dépôt des candidatures à la Présidence serait fixé au vendredi 10 mai, à midi. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française et sur celles du projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française sont parvenues à l'adoption d'un texte commun. la demande du groupe Les Républicains, les explications de vote et le vote sur la proposition de loi tendant à renforcer les pouvoirs de police du maire dans la lutte contre l'introduction et la propagation des espèces toxiques envahissantes,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

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi n° 215, présentée par notre collègue Agnès Canayer, vise à renforcer les pouvoirs de police du maire dans la lutte contre l'introduction et la propagation des espèces toxiques envahissantes. Cette proposition de loi tend plus spécifiquement à donner des pouvoirs au maire, afin qu'il puisse lutter contre les frelons asiatiques. Les maires sont en effet régulièrement interpellés par leurs administrés, qui, inquiets, scrutent et détectent un nid sur leur propriété, sur des espaces privés voisins ou même sur des espaces publics. Ils n'ont cependant aucune compétence lorsque le nid est situé sur une propriété privée dont le propriétaire refuse de donner l'autorisation de pénétrer ou d'agir, sauf s'il existe une menace grave et imminente pour la sécurité publique. Je commencerai mon intervention par une rapide présentation des espèces exotiques envahissantes. L'introduction de nouvelles espèces sur le territoire national n'est pas un phénomène récent. Avec le développement des échanges au niveau mondial, il s'est toutefois accéléré et de nombreuses espèces végétales ou animales arrivent sur le sol national. Au total, 14 000 sont comptabilisées.

Certaines ont un impact écologique, avec la création de désordres au niveau de l'écosystème faunique et floral : elles représentent ainsi la troisième menace pour la biodiversité à l'échelon mondial. D'autres ont un impact économique, avec une menace sur l'agriculture, par exemple, ou sanitaire, avec une menace pour la santé publique, comme c'est le cas de l'ambroisie à feuilles d'armoise, qui provoque des allergies. Les pouvoirs publics se sont rapidement rendu compte de la nécessité de coordonner au plus haut niveau la lutte contre ces espèces. Une convention internationale a tout d'abord été signée en 1992, avant que le sujet ne soit appréhendé à l'échelon européen en 2004. La notion d'espèces exotiques envahissantes a fait son apparition dans le droit national en 2016. La lutte contre les espèces exotiques envahissantes n'est efficace qu'au début de leur implantation sur le territoire. À ce moment-là, une opération rapide peut permettre d'éradiquer les spécimens d'une espèce sur le territoire à moindre coût. Après cela, l'espèce s'est diffusée et la stratégie de lutte doit s'orienter vers une gestion de la population globale et une protection des espèces autochtones qu'elle menace. Cette stratégie est alors beaucoup plus coûteuse. En France, c'est le préfet qui dispose du pouvoir de police pour lutter contre l'introduction et la propagation de ces espèces : il peut notamment intervenir à ce titre sur les propriétés privées. En cas de menace grave et imminente pour la santé publique et la sécurité, le maire peut également prendre, à défaut des propriétaires, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette menace au titre de son pouvoir de police générale ; c'est l'article L. 2212-4 du code général des collectivités Il peut, dans ce cadre, ordonner la destruction de certaines espèces exotiques envahissantes. Mais revenons plus précisément au frelon asiatique. Une seule reine frelon asiatique a été introduite en France en 2004 à l'intérieur de poteries importées de Chine. Présent dans treize départements en 2006, le frelon asiatique avait envahi cinquante-six départements en 2012 et a depuis conquis la France métropolitaine entière, à l'exception de la Corse. Le cycle de vie des frelons asiatiques est annuel. Les reines sortent de l'hibernation au printemps et fondent de nouveaux nids. Pendant l'été, les frelons chassent les insectes pour nourrir leurs larves, surtout les abeilles et les guêpes. Puis, la colonie meurt naturellement en hiver. Seules les femelles fécondées survivent en se protégeant du froid. Ils ne reviennent jamais dans le nid de l'année précédente ; il faut le savoir. piqûre n'est pas plus dangereuse pour l'homme que la piqûre du frelon européen ou que celle des guêpes. En revanche, les frelons asiatiques représentent un vrai danger pour les abeilles domestiques, donc pour l'apiculture. La stratégie d'éradication des nids n'est pas très efficace et coûte actuellement très cher. Nous ne constatons aucune diminution du nombre de frelons asiatiques. Au vu de la vitesse de propagation de l'espèce, il semble aujourd'hui que son éradication soit, sinon impossible, du moins très difficile. La recherche se concentre alors sur la protection des ruches. Le frelon asiatique est classé parmi les espèces exotiques envahissantes et les dangers sanitaires. Le pouvoir de police spéciale en la matière appartient donc au préfet. au préfet. Cependant, au titre de son pouvoir de police générale, le maire peut intervenir en cas de menace grave et imminente pour la sécurité publique. Je me suis attaché à décrire dans mon rapport les possibilités dont disposent les maires pour lutter contre le frelon asiatique et pour répondre aux sollicitations de leurs administrés en la matière. La proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui vise à donner de nouveaux pouvoirs au maire dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Lesquels ? L'auteur de la proposition envisageait initialement de permettre au maire de mettre en demeure le propriétaire d'agir contre les espèces exotiques envahissantes présentes sur sa propriété et, à défaut, de procéder à l'exécution de ces opérations aux frais du propriétaire. Plusieurs effets indésirables étaient toutefois à craindre : l'erreur sur l'identification des espèces, le maire n'étant pas systématiquement un biologiste l'emploi des techniques de lutte et les moyens utilisés sans encadrement, ce qui pourrait porter atteinte à la biodiversité au lieu de la protéger ; un risque de mise en cause de la responsabilité du maire en cas de mauvaises actions ou d'inaction la concurrence des pouvoirs de police avec le préfet, susceptible de conduire à la déresponsabilisation des deux autorités. En outre, mettre ces opérations à la charge du propriétaire pourrait avoir un impact négatif en matière de suivi scientifique de la diffusion de l'espèce, avec une diminution des signalements. Un nouveau pouvoir de police spéciale augmenterait les risques de contentieux, ce qui rendrait encore plus difficile l'exercice du mandat, en particulier pour les petites communes qui ne disposent pas de service juridique. Ce dernier point nous a notamment été souligné par Après avoir évalué les différentes hypothèses, la commission des lois a choisi, dans le cadre de la procédure de législation en commission, une autre solution. Celle-ci consiste, d'une part, à rappeler aux maires les pouvoirs dont ils disposent en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, en particulier les frelons asiatiques, et, d'autre part, à consacrer la possibilité pour les maires de saisir le préfet du département lorsqu'ils détectent des espèces exotiques envahissantes sur le territoire communal. Une telle position responsabilise les préfets en leur permettant de prendre les mesures pertinentes à la suite de ce signalement. Le maire aura un rôle de facilitateur et de sentinelle dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Il pourra ainsi sensibiliser et informer le public sur les risques. Il pourra jouer le rôle d'intermédiaire pour permettre une action sur les propriétés privées. Il formera un maillon essentiel de la chaîne de détection précoce des espèces, en opérant un signalement aux autorités chargées de la lutte. La Merci,

Mais je voulais faire un rappel au règlement fondé, notamment, sur l'article 34 de la Constitution. En effet, le texte tel qu'il nous est présenté a cette particularité d'être totalement inutile, puisqu'il prévoit simplement que le maire peut téléphoner ou écrire au préfet s'il est avisé de l'existence d'insectes toxiques sur le territoire de sa commune.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs,

un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, notamment 40 % des amphibiens, 33 % des récifs coralliens et 33 % des mammifères marins. Le rapport isole des causes et propose des pistes d'action. Cinq causes principales sont évoquées. La première est l'artificialisation et la fragmentation des milieux. La deuxième est la surexploitation des ressources naturelles. La troisième est le changement climatique. La quatrième, ce sont les pollutions. Et les espèces exotiques envahissantes dont nous parlons aujourd'hui sont la cinquième cause d'extinction ou de réduction de la biodiversité dans le monde.

hier et avant-hier. Cela a donné lieu à la première adoption d'une charte mondiale pour la biodiversité, signée par tous les membres du G7 et par les pays de différents continents

envahissantes sont originaires d'autres continents. Elles ont été introduites par l'homme, volontairement ou parfois accidentellement, comme c'est très probablement le cas, vous l'avez rappelé, s'agissant du frelon asiatique. Ce phénomène a pris une ampleur considérable depuis la Révolution industrielle, avec l'augmentation des flux de passagers et de marchandises à travers le monde.

Ces espèces sont à l'origine d'impacts négatifs multiples : des impacts environnementaux, des impacts économiques sur l'agriculture, sur le tourisme, et des impacts sanitaires sur la santé humaine. Mais ces espèces ont un impact particulièrement important dans nos outre-mer. Je le rappelle, nos outre-mer recèlent environ 80 % de la biodiversité française. Or cette biodiversité est spécifique et fragile. Elle est soumise à des flux importants, qui peuvent être autant de vecteurs de propagation. Les espèces exotiques envahissantes sont donc un problème sanitaire au sens large, avec un impact sur la santé de l'environnement, la santé vétérinaire, la santé des végétaux et la santé humaine. Du coup, plus ces espèces sont détectées précocement, meilleures sont les chances de parvenir à leur éradication dans un court laps de temps. En effet, lorsque le phénomène devient visible, il est souvent trop tard pour agir, et la détection dépend bien souvent de notre capacité collective à arpenter la nature et à sillonner le territoire, les techniques de lutte empiriques apparaissant parfois comme totalement dépassées. Certaines espèces- c'est le cas du frelon asiatique -sont trop largement répandues pour pouvoir être facilement éradiquées. l'échelon international, la Convention pour la diversité biologique intègre dans son programme stratégique 2011-2020, qui s'appelle l'agenda d'Aichi, un objectif spécifique sur ces espèces exotiques envahissantes. C'est d'ailleurs l'un des 4 objectifs sur 20 sur sur lesquels le rapport relatif à la biodiversité dont je parlais constate que des progrès satisfaisants ont été réalisés. En 2014, l'Europe a édicté un règlement qui liste les espèces et qui pose des interdictions sur ces espèces : interdiction de détention, de transport, d'utilisation, etc. la France s'est dotée, au travers de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, d'outils permettant de contrôler l'introduction sur notre territoire ou dans le milieu naturel, ainsi que la détention, le transport et l'utilisation de ces espèces. Cette réglementation nationale relève à la fois du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, du ministère de la santé et du ministère de la transition écologique et solidaire. La problématique monte donc en puissance. Il me semble important que le Sénat s'en saisisse. C'est un sujet du quotidien pour nos concitoyens. Cela nécessite une coordination forte entre les acteurs de terrain impliqués à différentes échelles géographiques et la concentration de la lutte sur les espaces et sur les espèces prioritaires, car il n'est pas possible de vouloir agir sur tous les fronts. a présenté la problématique du frelon asiatique sur la base d'une proposition de loi proposée par Mme Agnès Canayer. Ce texte confiait au maire un pouvoir de police renforcé pouvant exiger du propriétaire une action de lutte contre les espèces exotiques envahissantes présentes sur sa propriété. comme vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, cette proposition de loi soulevait différentes questions, notamment des risques d'erreur d'appréciation, de traitement inapproprié, de dispersion des moyens, qui ne conduisent pas forcément à l'efficacité recherchée en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Le maire peut et doit jouer un rôle de sentinelle, d'informateur à l'égard de ses administrés sur cette problématique. C'est le sens de l'amendement de M. le rapporteur, sur lequel le Gouvernement a émis un avis favorable ; il a été adopté par la commission. commission. À ce jour, il n'existe aucune solution totalement efficace de lutte contre le frelon asiatique. Les pièges physiques ne sont pas sélectifs et les biocides conduisent parfois à des pollutions diffuses. Il est préférable, comme vous l'avez rappelé, de se concentrer sur la protection des ruches par encagement. des ruches par encagement. L'espèce ne présente pas de danger pour l'homme, du moins pas plus que les espèces locales. Le grand opérateur issu de la fusion de l'Agence française de la biodiversité, l'AFB, et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à savoir l'Office français de la biodiversité, sera un acteur de premier plan, à l'appui des maires et des préfets sur la problématique des espèces exotiques envahissantes. Ses deux composantes travaillent déjà activement sur le sujet en matière de gestion, de prévention, de formation des gestionnaires et de communication. En liaison avec la stratégie nationale dont je parlais, un Centre de ressources national sur les espèces exotiques envahissantes a d'ores et déjà été créé auprès de l'AFB, animé avec le Comité français des associations de la nature. Ce centre fournit des informations sur les espèces présentes sur le territoire métropolitain, mais aussi en outre-mer, sur les techniques de gestion, sur la réglementation. Il produit une lettre d'information transmise régulièrement à plus de 1 500 acteurs de terrain. acteurs de terrain. La France dispose déjà de beaucoup des outils nécessaires pour une lutte efficace, ciblée, à travers une chaîne de décision opérationnelle et une mobilisation des acteurs locaux.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes appelés à voter cet après-midi vise à renforcer la lutte contre la propagation d'espèces exotiques envahissantes. En effet, l'introduction volontaire ou fortuite d'espèces exotiques envahissantes est l'une des premières causes majeures d'atteinte à la biodiversité dans nos territoires. Sorties de leur milieu naturel et introduites dans le nôtre, ces espèces déséquilibrent les écosystèmes. De par sa position de carrefour géographique, le territoire métropolitain est fortement touché par ces espèces, ce qui entraîne des dommages sanitaires et économiques considérables, notamment dans les filières agricoles et forestières. En effet, n'ayant plus à craindre leurs prédateurs naturels, elles croissent démesurément et menacent, voire détruisent, les espèces qui préexistaient. C'est le cas- cela a été rappelé -du frelon asiatique, qui parasite les ruchers en se nourrissant des abeilles. C'est également le cas du ver, dont la le cas du ver, dont la proie est le lombric. Face à ce danger, il faut donc prévenir l'introduction de telles espèces, mais il faut surtout agir rapidement lorsque l'introduction n'a pu être empêchée, et pour que celle-ci ne devienne pas invasive. 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le préfet a le pouvoir de procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite. C'est pourquoi il est important que l'État puisse agir afin de préserver la biodiversité de nos territoires, mais aussi la santé de nos concitoyens. La proposition de loi que nous nous apprêtons à voter aujourd'hui met en lumière le fait que le dispositif existant n'est pas suffisant et doit être complété. Elle vise à conférer au maire le pouvoir d'avertir l'autorité administrative compétente lorsqu'il constate la présence dans le milieu naturel d'une ou plusieurs espèces exotiques envahissantes. maire est trop souvent démuni face aux sollicitations de ses administrés, il nous semble préférable qu'il relaie l'information au préfet, afin que celui-ci se charge de déterminer les actions à entreprendre. Car identifier l'espèce en cause et déterminer l'action idoine requièrent une certaine expertise que ne détient pas nécessairement le maire. De plus, il est important que les opérations de lutte contre les espèces exotiques envahissantes conservent un financement public. Dans la mesure où la propagation de ces espèces menace et met en danger des écosystèmes de l'ensemble de nos territoires, le sujet relève de l'intérêt général. Nous sommes tous concernés par les externalités négatives de ces espèces et de leur propagation. C'est pourquoi, même si le groupe Les Indépendants est défavorable à l'augmentation des dépenses publiques, il nous paraît juste que de telles opérations restent financées par la puissance publique. Les spécimens de ces espèces n'ont que faire des frontières administratives de notre territoire. C'est par conséquent à l'État qu'il revient de mener et de coordonner la lutte. À l'heure où nous connaissons la sixième extinction animale de masse, l'enjeu est majeur et le temps presse. Nous devons tous avoir comme objectif la plus grande efficacité. Seule une politique nationale pourra apporter une solution à la mesure de la situation. Le groupe Les Indépendants soutient l'objectif de cette proposition de loi. Nous sommes cependant convaincus qu'une telle mesure devra s'accompagner d'autres actions en faveur de la préservation de nos écosystèmes si nous voulons sauvegarder la biodiversité de nos territoires. La parole

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,

En revanche, d'autres espèces exotiques envahissantes, qu'elles soient animales ou végétales, impactent particulièrement les territoires ultramarins, qui, rappelons-le, comme l'a dit Mme la secrétaire d'État, Je pense notamment à la liane papillon à La Réunion, à la tourterelle turque en Guadeloupe, au rat noir dans différentes îles, à l'iguane vert en Martinique et en Guadeloupe ou à la vigne marronne à Mayotte. La lutte contre ces espèces constitue donc un défi croissant pour préserver les richesses naturelles exceptionnelles de ces territoires. Motivée par l'expansion continue du frelon asiatique sur l'ensemble du territoire hexagonal, la proposition de loi, qui nous a été soumise en procédure de législation en commission, visait de façon plus générale à renforcer les pouvoirs de police des maires dans la lutte contre l'introduction et la propagation de ces espèces exotiques envahissantes, en lui permettant de mettre en demeure le propriétaire d'un terrain où s'est implantée une de ces espèces, de faire procéder à leur capture, à leur prélèvement, à leur garde ou à leur destruction. Si ledit propriétaire n'obtempérait pas dans le délai fixé par le maire, les dispositions du texte autorisaient celui-ci à agir en ses lieu, place et frais. Conscient que cette proposition de loi répond à une véritable préoccupation de nos concitoyens, qui interpellent très régulièrement leur maire, elle nous paraissait néanmoins comporter en sa rédaction initiale de nombreux effets indésirables, comme le soulignait M. le rapporteur. En effet, outre le fait que les maires disposent déjà de moyens au titre de leur pouvoir de police générale pour lutter contre les frelons asiatiques et autres « fléaux calamiteux » en cas de danger grave et imminent, le présent texte aurait pu entraîner des conséquences fâcheuses en matière de responsabilité. Nous savons que le but recherché par les auteurs de cette proposition de loi n'est pas de rendre l'exercice du mandat de maire plus difficile qu'il ne l'est aujourd'hui et qu'il s'agit bien au contraire de le faciliter. Par ailleurs, la lutte contre les espèces toxiques envahissantes nécessite des compétences naturalistes et techniques sans lesquelles les interventions sont au mieux inefficaces, au pire dangereuses pour l'environnement- en raison, par exemple, de l'emploi de produits inadaptés et toxiques -et pour la biodiversité- en cas d'erreur sur l'identification des espèces. En outre, faire peser le coût des interventions sur les particuliers, pourrait avoir comme conséquence la diminution des signalements de ces espèces aux scientifiques et aux pouvoirs publics. C'est la raison pour laquelle le texte issu de notre commission, qui rappelle aux maires les pouvoirs dont ils disposent aujourd'hui en la matière et leur consacre un rôle d'alerte auprès du préfet lorsqu'ils constatent la présence de spécimens sur le territoire communal, nous satisfait. La discussion autour de cette proposition de loi a eu le mérite de poser et de clarifier la question de l'articulation adéquate entre les pouvoirs du préfet et ceux des maires. Elle a Elle a également permis d'évoquer la prise en charge du coût de ces interventions. Le groupe La République En Marche se ralliera donc à la position de compromis retenue par le rapporteur et votera en faveur de la proposition de loi ainsi modifiée.

Le texte soumis à notre approbation améliore incontestablement la proposition initiale, qui, au final, chargeait les maires, qui n'en manquent déjà pas, d'obligations et de responsabilités nouvelles non seulement en matière sanitaire, mais aussi en matière En l'absence de mise en oeuvre de la procédure prévue, la commune devant faire l'avance des frais sans certitude d'être remboursée par le contrevenant, le maire et la commune auraient pu être mis en cause en cas d'accident dû à l'un de ces hyménoptères malvenus. Mieux vaut donc laisser cette charge, comme le prévoit d'ailleurs la loi, au préfet et aux spécialistes de la « petite bête », qui peuplent les Le texte de la commission évite cet écueil, mais vise-t-il à ajouter un outil de lutte, dont nous ne disposerions pas, contre les espèces invasives ? Évidemment non, ... puisque tout élu municipal, voire tout citoyen, peut déjà aviser l'autorité administrative des dangers potentiels dont il aurait connaissance. Absolument ! C'est même là le devoir de tout On l'aura compris, le groupe CRCE s'abstiendra d'ajouter une nouvelle disposition superfétatoire à toutes celles qui existent déjà.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les espèces exotiques envahissantes ont des effets délétères en matière de biodiversité mondiale, de risques économiques pour les territoires impactés et de santé publique. Parmi ces dernières, le frelon asiatique en est l'un des spécimens les plus redoutables. Identifié pour la première fois en France il y a une quinzaine d'années après son importation involontaire, il s'est très rapidement propagé sur le territoire et est désormais installé dans toute la France métropolitaine, à l'exception de la Corse. Le frelon asiatique est responsable de dégâts considérables dans les lieux où il sévit. Il s'attaque aux abeilles et aux ruches, causant l'anéantissement de nombreuses colonies. Cette surmortalité est source de fortes inquiétudes, les abeilles étant, en tant qu'insectes pollinisateurs, un maillon essentiel de notre écosystème. Ma collègue Nicole Bonnefoy, impliquée de longue date sur ce sujet, a ainsi déposé dès 2011 une proposition de loi tendant à créer un fonds de prévention contre la prolifération du frelon asiatique, notre groupe politique s'est mobilisé à plusieurs reprises. Il faut également le rappeler, la piqûre du frelon asiatique peut s'avérer potentiellement mortelle pour l'homme et la présence d'un nid constitue une vraie menace pour les particuliers. La lutte contre cette espèce nuisible repose aujourd'hui essentiellement sur la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L'article L. 411-6 du code de l'environnement prévoit ainsi que sont interdits l'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant d'espèces exotiques envahissantes. L'arrêté ministériel du 14 février 2018 inclut le frelon asiatique dans la liste de ces espèces. S'agissant des opérations de lutte, elles sont prévues par l'article L. 411-8 du même code, qui dispose que l'autorité administrative, dès le constat de la présence d'une des espèces mentionnées dans l'arrêté, peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens. L'article R. 411-46 désigne enfin le préfet de département comme autorité administrative compétente. Le déploiement du frelon asiatique sur l'ensemble du territoire et sa persistance nécessitent de mettre en oeuvre des mesures à grande échelle, les actions localisées paraissant insuffisantes à enrayer sa prolifération. Une stratégie nationale de lutte, telle que celle qui est prévue par le code de l'environnement, semble donc aujourd'hui incontournable. Pourtant, en réponse à plusieurs questions adressées par des sénateurs, le Gouvernement reconnaît « qu'il n'y a actuellement aucune stratégie collective reconnue efficace Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a, quant à lui, annoncé avoir décidé de subventionner des actions de recherche visant à valider des méthodes de lutte sur le plan de leur efficacité et de leur innocuité sur l'environnement. Il serait à cet égard utile, madame la secrétaire d'État, que le Gouvernement puisse nous informer de l'avancée de ces recherches. En tout état de cause, les travaux de notre commission des lois, réunie jeudi dernier pour examiner la proposition de loi de notre collègue Agnès Canayer, me paraissent aller dans le bon sens puisqu'ils clarifient le rôle du maire en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Il faut, à cet égard, rappeler que, en l'état actuel du droit et au titre de son pouvoir de police générale, celui-ci peut déjà intervenir sur les propriétés privées en cas de danger grave et imminent pour la sécurité publique, en complémentarité avec le pouvoir de police spéciale du préfet. Notre commission a, en outre, décidé de consacrer dans la loi le pouvoir d'alerte du maire auprès du préfet lorsqu'il constate la présence d'une de ces espèces sur le territoire communal afin que ce dernier puisse prendre les mesures nécessaires à la suite d'un tel signalement, ce qui n'est, en fait, Nous avons enfin choisi de valoriser le rôle d'intermédiaire du maire, afin de sensibiliser les citoyens aux risques que constituent ces espèces exotiques envahissantes et d'obtenir l'accord des administrés pour qu'une intervention sur leur propriété privée soit mise en oeuvre. Sur ce sujet, j'ai rappelé la nécessité de ne pas imputer aux particuliers les frais relatifs à ces opérations, afin d'éviter que ceux-ci ne décident, pour éviter ces coûts, de procéder eux-mêmes à la destruction des nids de frelons au travers de manoeuvres hasardeuses, voire dangereuses. La proposition de loi ainsi modifiée nous paraît adaptée et équilibrée. Elle permettra, nous l'espérons, d'aboutir à une lutte plus efficace contre ces espèces exotiques envahissantes. Notre groupe politique votera donc en faveur de ce texte. Bravo pour votre

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques révèle une augmentation d'environ 70 % du nombre d'espèces exotiques envahissantes depuis 1970 dans 21 pays. Ces espèces contribuent au déclin de notre biodiversité, y compris par leur impact sur l'agriculture. Parmi ces espèces, le frelon asiatique pose de véritables difficultés dans tous nos territoires du fait de sa prédation à l'encontre des colonies d'abeilles domestiques, alors que ces dernières subissent les effets du changement climatique et de certains pesticides. Répondant aux préoccupations de nos concitoyens et des élus, les auteurs de la proposition de loi ont souhaité renforcer les pouvoirs du maire en lui permettant d'intervenir contre ces espèces, au sein des propriétés privées et aux frais du propriétaire. Bien que comprenant parfaitement la frustration de certains maires de ne pas pouvoir intervenir systématiquement en l'absence d'accord du propriétaire- cela m'est arrivé lorsque j'étais maire -, le dispositif proposé ne nous semblait pas le mieux adapté pour freiner l'expansion de l'espèce. outre les conséquences juridiques fâcheuses qu'il aurait pu engendrer en ouvrant la porte à la mise en cause de la responsabilité des maires, il aurait eu pour résultat de dissuader les propriétaires de signaler les nids et de les inciter à les détruire, à leurs risques et périls. Or nous avons besoin d'une connaissance la plus exacte possible de l'espèce et de méthodes de destruction sélectives et moins nocives pour l'environnement. De surcroît, la reconnaissance des espèces ne va pas toujours de soi, le frelon asiatique pouvant être confondu avec le frelon d'Europe, la guêpe des buissons, la scolie des jardins et autres Ces remarques sont applicables à l'ensemble des espèces exotiques envahissantes. Désormais le texte, tel qu'il résulte des travaux en commission, est dénué de portée normative. Lorsqu'il est saisi de la présence de ces espèces, le maire s'adresse d'ores et déjà au préfet, sans que la loi l'y oblige. Son rôle consacré dans la loi ne serait que celui de « pouvoir » aviser le préfet, qui, en vertu de l'article L. 411-8 du code de l'environnement, peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens, y compris sur les propriétés privées. Mes chers collègues, il n'est nul besoin de rappeler au maire qu'il dispose de son pouvoir de police générale.

En l'absence de prise en charge financière par l'État, le coeur du problème réside dans la réponse à géométrie variable qu'obtiennent nos concitoyens, qui ne sont pas sur un pied d'égalité selon que la collectivité territoriale participe ou non au coût de la destruction. Nous concevons que l'intention des auteurs de la proposition de loi soit de consacrer le rôle d'alerte du maire, mais il eût été plus pertinent de renforcer les obligations du préfet en la matière, car le problème reste entier, le préfet décidant des suites à donner selon son bon vouloir. La problématique des espèces exotiques envahissantes devenant dans le cas du frelon asiatique une menace de caractère national, la responsabilité de l'État est d'aboutir à l'élaboration d'un système de prévention et d'intervention plus réactif, car, une fois que ces espèces sont installées, il est souvent trop tard. Le frelon asiatique,

Mes chers collègues, il faut agir de manière prudente et une stratégie nationale doit être mise en place pour accompagner les particuliers, les professionnels et les collectivités territoriales dans la destruction des nids si cette solution est considérée comme indispensable. En tout état de cause, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ne peut uniquement être abordée par le seul prisme de la destruction, mais elle doit faire l'objet d'une recherche à rétablir les équilibres écologiques, car les interventions peuvent se retourner contre nos espèces domestiques. En conclusion, le groupe du RDSE votera ce texte, même modifié et vidé de ses contraintes et de son caractère normatif. effet, comme auraient pu l'affirmer les jésuites-et c'est un radical qui le dit ! -, l'intention dans ce cas vaut l'action

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous terminons aujourd'hui l'étude de la proposition de loi tendant à renforcer les pouvoirs de police du maire dans la lutte contre l'introduction et la propagation des espèces toxiques envahissantes, dont nous avons examiné jeudi dernier les articles grâce à la procédure de législation en commission. Comme Comme je l'ai déjà dit à cette occasion, lorsque j'ai découvert le programme de la commission des lois, j'ai commencé par me dire qu'il y avait erreur d'aiguillage : pour quelle raison le frelon asiatique s'invitait-il en discussion devant la commission des lois ? Lors de l'examen en commission jeudi, les diverses interventions de mes collègues, tous confrontés à ce problème, m'ont un peu éclairé. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles m'ont convaincu de l'intérêt de légiférer sur le sujet. Le maire est

Un débat sur le sujet n'était sans doute pas inutile pour clarifier les compétences du maire et rappeler l'importance du rôle des préfets en la matière, mais pas suffisamment pour aboutir à la nécessité d'adopter une nouvelle loi. Si les travaux de la commission ont pu clarifier l'articulation des pouvoirs respectifs du maire et du préfet, et donner aux maires ce que j'appellerai un « mode d'emploi » face aux frelons asiatiques et aux espèces envahissantes, je m'en réjouis évidemment.

d'avril 2019 : « Le juge rappelle qu'il appartient au maire d'une commune, en vertu de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Les interdictions édictées à ce titre ne doivent être ni générales ni absolues, et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu'il s'agit de prévenir. Ces mesures de police doivent être strictement proportionnées à leur nécessité. d'un arrêt du 9 juillet dernier de la cour administrative de Marseille concernant la commune de Beaucaire, qui était confrontée à ce même type de problèmes. que les maires n'ont pas besoin d'une nouvelle législation pour intervenir, avec les services compétents de l'État, dans la lutte contre l'introduction et la propagation des espèces toxiques envahissantes. La population française serait d'ailleurs certainement moins nombreuse si les maires n'étaient pas n'étaient pas intervenus les fois précédentes ! Cependant, ce texte aura sans doute le mérite de sensibiliser les pouvoirs publics et les maires sur ces questions. S'agissant de notre vote, le groupe Union Centriste s'abstiendra sur cette proposition de loi. La

des espèces exotiques envahissantes, et tout particulièrement du frelon asiatique. Comme pour beaucoup de sujets, les maires sont les premiers réceptacles de l'anxiété de leurs administrés. Ils sont notamment sollicités sans avoir les moyens scientifiques, juridiques et matériels de répondre à leurs demandes. C'est pourquoi je salue l'initiative de notre collègue Agnès Canayer, qui nous permet de faire le point sur ce sujet et d'apporter une réponse pragmatique à une préoccupation bien réelle. Je salue également l'excellent travail de notre collègue rapporteur, Vincent Segouin. Ce texte est attendu par les maires et le Sénat est dans son rôle lorsqu'il cherche des solutions adaptées aux collectivités territoriales. C'est bien vrai ! Je pense, notamment, aux maires de petites communes, que je rencontre, qui se sentent démunis face à la demande de leurs concitoyens ayant détecté des nids de frelons sur leur propriété ou sur celle de leur voisin. Cela pourrait paraître anecdotique, mais c'est une réalité vécue au quotidien dans nos mairies. Si certaines espèces exotiques n'ont aucune incidence, d'autres, qualifiées d'envahissantes, ont des impacts importants sur la biodiversité, l'économie et la santé. La lutte contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes participe à la préservation de la biodiversité, en grand danger comme le démontre le rapport rendu hier à l'Unesco par les experts de l'IPBES. À ce titre, le frelon asiatique est un bon exemple. Arrivé en France en 2004, il s'est répandu, en une quinzaine d'années, sur l'ensemble des départements français. Il constitue une réelle menace pour de nombreuses espèces d'insectes, tout particulièrement pour les abeilles domestiques. C'est pourquoi, depuis un arrêté du 26 décembre 2012, le frelon est classé dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie, pour l'abeille domestique, sur tout le territoire national. En France, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a donné une définition des espèces exotiques envahissantes. La même loi confie aux représentants de l'État, les préfets, la compétence de lutter contre l'introduction et la prolifération de ces espèces. Il leur revient donc de prendre les mesures adéquates en vertu de leur pouvoir de police spéciale. Toutefois, ils semblent avoir, suivant les départements, une vision différente de l'exercice de leurs prérogatives. Quant aux élus locaux, certains ont fait le choix de prendre en charge, au niveau communal ou intercommunal, la destruction des nids de frelons chez les particuliers ou ils fournissent des pièges. Souvent, ils diffusent de l'information auprès de leurs administrés sur l'attitude à adopter en cas de découverte de nids de frelons. Dans sa version initiale, la proposition de loi tendait à renforcer les pouvoirs de police du maire dans la lutte contre l'introduction et la prolifération de ces espèces. Il était ainsi prévu de permettre aux maires, en cas de présence sur une propriété privée d'une espèce exotique envahissante, négligent de faire procéder à sa capture, à son prélèvement, à sa garde ou à sa destruction. Dans l'hypothèse où le propriétaire n'obtempère pas à la mise en demeure, après un certain délai, le maire peut faire procéder d'office à l'exécution de ces opérations, aux frais du propriétaire. Il s'agissait de créer un pouvoir de police spéciale pour les maires. Toutefois, cette proposition a paru poser des inconvénients juridiques, environnementaux et matériels. En effet, la coexistence de deux pouvoirs de police spéciale risquait de conduire à une déresponsabilisation. L'efficacité passe par une clarification du rôle de chacun. De plus, il est toujours délicat pour une commune d'intervenir sur une propriété privée. La probabilité d'un contentieux est forte. C'est pourquoi la proposition de la commission des lois visant à compléter l'article L. 411-8 du code de l'environnement, en laissant aux préfets, seuls, la compétence de lutter contre l'introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes et à faire du maire un lanceur d'alerte me paraît un bon compromis. Dans la version adoptée en commission, le maire devient donc un maillon essentiel dans la chaîne de lutte contre ces espèces. Véritable sentinelle, il aura pour mission d'informer la population sur les risques et pourra alerter le préfet en cas de découverte d'espèces envahissantes sur sa commune, pour permettre de prendre les mesures adéquates. En cas de menace grave et imminente, le maire a toujours la possibilité d'agir en vertu de son pouvoir de police générale. Cette proposition de loi est examinée suivant la procédure de législation en commission, mise en place au Sénat sur l'initiative de son président, Gérard Larcher.

a pour objet de renforcer l'intervention du maire dans la lutte contre l'introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes, et tout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

sur la réforme de la politique agricole commune, présentée par M. Daniel Gremillet, Mme Pascale Gruny, MM. Claude Haut et Franck Montaugé

nous nous apprêtons aujourd'hui à débattre d'une troisième proposition de résolution européenne du Sénat consacrée à la prochaine réforme de la politique agricole commune, Le Sénat a déjà adopté deux résolutions européennes à ce sujet, les 8 septembre 2017 et 6 juin 2018. Par cette nouvelle initiative, nous entendons indiquer au Gouvernement les préconisations de la Haute Assemblée et exprimer nos inquiétudes à l'égard des propositions formulées par la Commission européenne. Pour mémoire, ces propositions de la Commission s'articulent autour de cinq grands axes : un nouveau mode de mise en oeuvre de la PAC supposé favoriser la simplicité et l'efficacité, grâce à davantage de subsidiarité un meilleur ciblage des aides et leur plafonnement à 100 000 euros par exploitation ; un renforcement notable des ambitions environnementales ; la promotion de la recherche et des innovations technologiques enfin, une diminution du budget agricole, estimée par le Parlement européen à 15 % en termes réels pour la période 2021-2027, comparée à la période 2014-2020. Cette réduction représente, en fait, la matrice de l'ensemble de la réforme. Depuis leur présentation, le 1 juin 2018, ces propositions sont demeurées largement inchangées, dans un contexte où les négociations entre les États membres au sein du Conseil sont apparues longues et difficiles. Au regard de tous ces éléments et des positions prises par les autorités françaises, il nous a semblé indispensable de revenir sur le sujet. Cette troisième proposition de résolution européenne, qui a été adoptée par nos commissions des affaires économiques et des affaires européennes, confirme et prolonge nos réflexions antérieures. Nous voulons une PAC forte, rénovée et répondant aux attentes des agriculteurs. Dans cet objectif, notre proposition de résolution comporte 28 demandes et recommandations, visant à : obtenir un budget stable en euros constants sur la période 2021-2027 et réaffirmer les termes des précédentes résolutions du Sénat rappeler que la PAC doit demeurer une priorité stratégique pour l'Union européenne ; souligner le fort risque que le nouveau mode de mise en oeuvre ne remette en cause la substance même de la politique agricole commune mettre en garde contre les perspectives de distorsions de concurrence supplémentaires, de dumping social et environnemental et de pénalisation des producteurs les plus vertueux demander de nouvelles améliorations en matière d'adaptation des règles de concurrence ou d'intervention, au-delà des progrès apportés par le règlement « Omnibus » du 13 décembre 2017 saluer les avancées en matière d'aides aux jeunes agriculteurs, de nouvelle réserve de gestion des crises et de soutien accru à la recherche et à l'innovation. Fort heureusement, les négociations sur les contours de la future réforme de la PAC sont loin d'être finies. Par ailleurs, les autorités françaises ont affirmé le caractère « inacceptable » des propositions de la Commission européenne en matière budgétaire dans le prochain cadre financier pluriannuel. Pour autant, nos agriculteurs ont grand besoin d'être rassurés. Il en va de même pour la représentation nationale. Vous êtes d'ailleurs bien placé pour savoir, monsieur le ministre, que le sujet de la PAC nous tient tous particulièrement à coeur, au point de transcender largement nos différentes sensibilités politiques.

en complément de l'intervention de notre collègue Claude Haut, j'axerai mon propos sur la comparaison entre les propositions du Sénat et le schéma de réforme envisagé par la Commission européenne. Or, en l'état actuel des choses, disons-le clairement : l'écart entre les deux apparaît tout à fait considérable. Certes, ce schéma comporte plusieurs points positifs. Notre collègue vient de les saluer. Néanmoins, le contenu général des négociations en cours suscite un très vif sentiment de malaise, en raison tout à la fois des contraintes budgétaires, du manque d'ambition et des risques soulevés par les orientations de la Commission européenne. Plus précisément, ces orientations ne reprennent que très imparfaitement, voire contredisent, aussi bien les recommandations des deux premières résolutions du Sénat, de 2017 et 2018, que celles de notre nouvelle, et troisième, proposition de résolution européenne sur la PAC. Nous déplorons le projet de diminution drastique du budget : en termes réels, baisse de 12 % pour le premier pilier et de 28 % pour le second. S'y ajoutent l'incertitude pesant sur le nouveau mode de mise en oeuvre de la PAC, des interrogations sur les nouvelles ambitions environnementales, ainsi que la perspective d'un quasi-sur l'adaptation des règles de concurrence aux spécificités agricoles. En dernière analyse, le risque ultime de la réforme en gestation est même celui d'une renationalisation de la politique agricole. Depuis de nombreuses années, en effet, les pays de l'Union affichent des divergences de vues de plus en plus profondes sur la PAC. Par cette proposition d'un nouveau mode de mise en oeuvre, la Commission manifeste surtout l'intention de mettre un terme à son travail de médiation pour trouver une position commune, en laissant désormais la main largement aux États membres pour la gestion de leur politique agricole. Or les obligations réglementaires et les standards permettant d'assurer de bonnes conditions agricoles et environnementales, qui figurent dans l'annexe du projet de la Commission, deviendraient presque tous optionnels. Les distorsions de concurrence ne pourraient, dès lors, que s'accentuer dans une course au moins-disant environnemental conduite en toute légalité, au détriment des producteurs les plus vertueux, notamment français, alors même qu'ils éprouvent déjà de grandes difficultés à vivre dignement du fruit de leur travail. Au surplus, la présentation détaillée du dispositif, qui comprend 142 articles et plusieurs annexes, conduit à craindre un simple « transfert de bureaucratie » de l'Union européenne vers les États membres, dont les agriculteurs ne tireraient aucun bénéfice. En définitive, seule la Commission européenne semblerait y trouver intérêt ... Ce changement radical d'approche fait craindre un fort risque de « renationalisation rampante On peut ainsi redouter, à terme, c'est-à-dire à la fin des années 2020, d'aboutir à 27 politiques agricoles qui ne seraient plus communes en rien. Cela marquerait la fin de la PAC telle qu'elle a été conçue et appliquée depuis l'origine, en 1962.

ainsi que la ligne directrice qui sous-tend notre proposition de résolution, afin de conjurer pareille perspective. Depuis le 6 juin 2018, date de notre dernier débat en séance publique avec votre prédécesseur, monsieur le ministre, PAC ont continué à avancer, sans malheureusement que les orientations défendues par la Commission européenne soient fondamentalement remises en question, au sein du Conseil, par les États membres. Or, monsieur le ministre, il y a urgence, car, plus le temps passe, plus ces orientations risquent de s'imposer à la longue. Le Président de la République nous donne parfois l'impression de nous écouter à Paris, mais de tenir un discours inverse à Bruxelles. Pour peser face à nos partenaires, il faut une parole constante et une voix qui ne tremble pas. Disons-le franchement : si les autorités politiques françaises ne réagissent pas maintenant, en envoyant un signal politique particulièrement fort, il sera définitivement trop tard ! La parole La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur

À cette occasion, j'avais relevé le paradoxe temporel de la proposition de réforme administrative et financière de la PAC proposée par la Commission. Il peut se résumer ainsi : c'est justement à l'heure où l'on parle d'une Europe en crise que la Commission européenne a délibérément choisi de sacrifier sa politique la plus européenne et la plus intégrée. Cette situation n'a pas changé et il est important de le rappeler à la veille des élections européennes. Modifier ainsi la PAC serait plus qu'une faute : ce serait un véritable renoncement. Un renoncement à l'égard de femmes et d'hommes travaillant jour et nuit, avec passion, pour nourrir le continent. À l'heure où il est si faciled'obtenir des produits alimentaires importés de moindre qualité, comment peut-on justifier de telles coupes drastiques dans les budgets européens, lesquelles viennent saper la compétitivité de nos exploitations au détriment de la sécurité sanitaire du continent ? un renoncement au regard de l'ambition agroenvironnementale de l'agriculture européenne. Comment pourrait-on demander aux agriculteurs de faire beaucoup plus avec beaucoup moins ? un renoncement face à une ambition stratégique que tous les autres grands pays du monde ont bien comprise. La PAC semble une priorité déclinante pour l'Union européenne, alors qu'il en va bien autrement pour toutes les autres grandes puissances agricoles.

déjà largement en tête -de 39 % et le Brésil de 44 %. Et la Commission ambitionne d'accélérer la réduction avec une baisse de 15 % en euros constants du budget de la PAC dans le prochain cadre financier pluriannuel. Cela fait un an que la position de la Commission est connue. Le Gouvernement a toujours déclaré, en public, être contre ce budget. Or, depuis notre dernier débat, en juin dernier, rien n'a évolué. Les coupes sont toujours là, au même niveau que ce qui avait été annoncé. Ce renoncement, monsieur le ministre, c'est aussi celui du Gouvernement dans la négociation européenne. Quelques lueurs d'espoir sont apparues, notamment au sein de la commission de l'agriculture du Parlement européen, qui, bien que politiquement contrainte, a proposé quelques avancées. Je pense notamment à la pérennisation jusqu'en 2050 du système des autorisations de plantation de vigne, seul outil de gestion du potentiel de production au sein de la PAC. Mais le bilan reste très terne. Enfin, et c'est sûrement le plus grave, c'est un renoncement au regard de l'idée européenne en cette veille d'élections. Les auditions de notre groupe de suivi ont mis en évidence un sentiment, largement répandu dans le monde agricole, de perte de sens de la politique agricole commune. Or la PAC a rempli, depuis 1962, un rôle fondateur essentiel pour garantir une nourriture en quantité suffisante et d'une qualité exemplaire à l'ensemble de l'Union européenne. Comme aime à le dire le président de la commission des affaires européennes, Jean Bizet, c'est une politique ancienne, mais loin d'être une vieille politique. Elle est la clef d'entrée pour relever les principaux défis du XXIsiècle. La position du Sénat a toujours été très claire cette proposition de résolution, fruit d'un travail transpartisan, la réaffirme haut et fort. Pour nos deux commissions, l'agriculture garantit l'indépendance alimentaire du continent européen, tout comme elle veille à la sécurité sanitaire des consommateurs européens. Elle contribue à la vitalité de nos territoires ruraux. Sans elle, les mécanismes d'aide alimentaire ne seraient pas ce qu'ils sont. Elle permet une meilleure préservation de l'environnement grâce à ses externalités positives qui bénéficient à l'ensemble de la société. L'agriculture doit être notre priorité stratégique. C'est pourquoi aucune réforme de la politique agricole commune ne sera satisfaisante sans une préservation d'un budget, d'une ambition en euros pour la Votre responsabilité, monsieur le ministre, est désormais de lutter contre ce renoncement et de faire évoluer les choses. Après, il sera trop tard ! La parole est à M. Franck Montaugé, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,pour la troisième fois, nous interpellons le Gouvernement sur le devenir, très préoccupant selon nous, de la plus grande politique intégrée de l'histoire de l'Union européenne, la PAC, une politique qui a longtemps été la clef de voûte de toutes les institutions européennes. Pour l'essentiel, les inquiétudes et les propositions que nous formulions dans les deux résolutions précédentes persistent. Les voici en quelques mots : une vision stratégique faible dans un contexte international où l'indépendance et l'autosuffisance alimentaires deviennent des enjeux majeurs des protections amoindries pour les agriculteurs dont le travail n'est pas reconnu à sa juste valeur et qui sont de plus en plusconfrontés aux aléas sanitaires, économiques etenvironnementaux ; une insuffisante prise en compte des attentes de la société etdes consommateurs en matière de qualité et de sécuritésanitaires des aliments. Dans ce contexte,

avec plus de 10 % de perte de revenu direct pour les agriculteurs et près de 30 % pour de développement territorial. En sus des problèmes du programme Leader, le message en direction des acteurs des territoires déjà en difficulté- agriculteurs, maires, etc. -est ici très négatif. C'est pourtant l'épure qui résulte du nouveau contrat de financement pluriannuel. Vous nous direz, monsieur le ministre, comment, dans un tel contexte, l'effort qui est demandé aux agriculteurs en matière de conversion et de transition vers l'agroécologie sera rendu possible par le Gouvernement.

Certains territoires et leurs producteurs sont victimes de la nouvelle carte. Je vous renouvelle la proposition gersoise de mettre en oeuvre sur ces territoires une démarche expérimentale de PSE. Nous avons tous les éléments- scientifiques, économiques et juridiques -pour nous y engager. Et s'il fallait ne pas prendre sur les crédits de la PAC, nous vous proposons de rémunérer ces services sur les fonds Horizon Europe- 100 milliards d'euros prévus tout de même sur la période 2021-2027 -, voire sur les fonds LIFE. Les syndicats agricoles y sont prêts. Il faut y aller ! Je terminerai sur la question centrale de la gouvernance de la future PAC. Prenons garde, monsieur le ministre, que ce qui, sous couvert de subsidiarité, est présenté comme une simplification de la gestion de la PAC ne se traduise dans les faits par une concurrence accrue entre agricultures nationales. Dans l'état actuel des propositions, pour le moins floues, le risque de renationalisation de la PAC est pour nous réel. Si cette voie devait être engagée, les inconvénients pour la France pourraient à terme être plus importants que les avantages. Mesurons-le et tirons-en les conséquences politiques ! Pour notre part, nous en appelons plutôt à des mécanismes européens communs et plus souples de gestion. Je pense à la réserve de crise et à l'article 224 qui permet de déroger aux règles de la concurrence, à la mise à disposition des exploitants agricoles d'une boîte à outils de gestion des risques auxquels ils sont confrontés, à des normes identiques- c'est très important -s'appliquant à l'ensemble des agricultures européennes, au refus des produits d'importation qui ne respectent pas les standards de production européens, et donc à la création d'une structure de contrôle sanitaire européen. La PAC est à un tournant aussi important que celui de 1992, qui avait consisté à s'aligner progressivement sur les prix des marchés par réduction des aides. Depuis l'ouverture de cette période, l'agriculture française se porte-t-elle mieux ? de certains acteurs des filières, mais certainement pas des producteurs. Cet enjeu social apparaît insuffisamment pris en compte dans les orientations de la Commission. Notre agriculture a aussi reculé à l'exportation et la question de sa compétitivité est posée. C'est à l'aune de ces problématiques, en plaçant les paysans et les producteurs agroalimentaires au coeur du raisonnement, que nous construirons une nouvelle étape de l'agriculture répondant aux demandes de la société européenne et aux enjeux de l'agriculture française. Le commissaire Hogan avouait que « les principes de la future réforme sont déjà acquis ». Alors, pourquoi en discutons-nous ? Quelle est en définitive, monsieur le ministre, la stratégie du gouvernement français pour que les principes de la future PAC servent les intérêts des agriculteurs français ?

pour permettre ces évolutions. La mutation de l'agriculture aujourd'hui en France se fait comme jamais elle ne s'est faite. Il n'existe aucune autre filière économique de notre pays

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui appelés à nous prononcer sur la troisième proposition de résolution européenne émanant du groupe de suivi sur la PAC, sur la PAC, mis en place conjointement en 2016 par la commission des affaires européennes et celle des affaires économiques, dont je salue les rapporteurs. Les deux précédentes PPRE ont été approuvées à l'unanimité par notre assemblée, respectivement en septembre 2017 et en juin 2018. Cette troisième proposition de résolution survient à un moment très particulier du calendrier. Nous sommes, en effet, à moins de trois semaines d'un scrutin européen très important, lequel définira les contours politiques du nouveau Parlement européen de Strasbourg qui, lui-même, déterminera les équilibres et les orientations de la future Commission européenne qui prendra officiellement ses fonctions le 1 novembre prochain. que M. Jean-Claude Juncker passera la main puisqu'il n'est pas candidat à sa succession. On sait aussi que, fort probablement, le Royaume-Uni aura choisi de quitter l'Union européenne à La Commission qui achève son mandat, comme toutes celles qui l'ont précédée, a fait l'objet de nombreuses critiques. Si certaines sont justifiées, je veux dire ici qu'il faut néanmoins rendre hommage à bon nombre de décisions et d'engagements pris par cette dernière, notamment au cours des deux dernières années. Le discours sur l'état de l'Union prononcé en septembre dernier par le président Juncker était particulièrement riche et offensif, insistant sur la nécessité pour l'Union d'affirmer sa souveraineté- on parle ici de souveraineté alimentaire -dans le cadre des valeurs fondatrices qui sont les siennes, à un moment où l'édifice européen est en proie à des menaces à peine voilées, tant à l'intérieur de son périmètre qu'à l'extérieur de celui-ci. Ce discours n'est pas sans faire écho à celui qui a été porté par le Président de la République française tout au long de sa campagne présidentielle et maintes fois réaffirmé depuis. Depuis deux ans, la Commission ainsi que les présidences successives du Conseil et les commissions du Parlement européen travaillent ardemment à la préparation du prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027, qui fixera les choix budgétaires de l'Union pour la prochaine mandature et même au-delà. La Commission, en dépit du Brexit qui occupe beaucoup ses services, a voulu aller vite pour tenter d'éviter les affres et parfois la confusion qui avaient régné- on s'en souvient ! -lors de la préparation

Cette volonté d'anticiper et d'accélérer le processus européen peut avoir ses bons côtés : ainsi, la réactivité accrue de l'Union quant à la production de directives sur des questions stratégiques stratégiques s'est largement améliorée par rapport à l'enlisement dont elle souffrait parfois dans le passé. Mais, dans le contexte particulier du prochain cadre financier pluriannuel, l'espoir de la Commission- heureusement déçu !-de le faire adopter en amont des échéances électorales de cette année avait quelque chose de très gênant d'un point de vue démocratique : en effet, une Commission et un Parlement sortants auraient, purement et simplement, défini par anticipation le cadre budgétaire de toute toute la mandature à venir, sans que les nouvelles instances concernées par celui-ci aient eu leur mot à dire. Si nous sommes parvenus à échapper à cette ineptie démocratique, la Commission sortante nous a cependant laissé un testament très directif et qui risque de peser lourd dans les négociations à venir. À sa décharge, il faut dire que le financement de l'Union européenne repose plus que jamais sur les contributions nationales des États membres, qui, rigueur budgétaire oblige, sont assez malthusiens quant aux moyens à allouer à l'Union et de plus en plus vigilants sur le taux de retour pour leur pays des investissements budgétaires. En contrepartie, les exigences de nouveaux investissements réclamés par tous dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la politique de la recherche et de l'innovation et pour développer Erasmus- j'en passe et des meilleurs

dites « classiques » et de TVA représentaient environ 80 % des ressources globales de l'Union, rendant plus facile l'allocation des dépenses pour les différentes politiques communautaires. Cela n'excuse évidemment pas les coupes importantes proposées par la Commission et soutenues par un certain nombre d'États quant au budget de la PAC pour la période 2021-2027, mais contribue quelque peu à les expliquer. Certes, il faut adapter et ajuster la PAC aux nouveaux défis de l'époque, comme cela a déjà été fait à de très multiples reprises depuis les années 1980. certaines des propositions de l'actuelle Commission pour le prochain cadre pluriannuel financier sont louables, comme le renforcement des aides aux jeunes agriculteurs, la volonté de consolider l'ambition environnementale et la recherche et l'innovation dans ce secteur, ainsi que la création d'une

fondateur de la PAC à sa création : celle de garantir la souveraineté alimentaire de l'Europe. La proposition de la Commission de consacrer 10 milliards d'euros, tirés du futur programme Horizon Europe, à la recherche et à l'innovation dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, du développement rural et de la bioéconomie, contre seulement 3,8 milliards d'euros dans l'actuel programme Horizon 2020, est certes une bonne chose. Ce qu'on appelle le, autrement dit l'agriculture de précision, peut apporter beaucoup à notre agriculture, tant en termes de qualité des produits que d'optimisation de la production, en ayant notamment

par la Commission ne sont pas encore suffisants et, en l'état, ces technologies appliquées à l'agriculture restent encore, pour diverses raisons, dont la formation et la connectivité du monde agricole, assez inaccessibles à près de 80 de nos agriculteurs. Pour toutes ces raisons et aussi pour toutes celles qui ont été rappelées par les rapporteurs, le groupe La République En Marche votera en faveur de cette proposition de résolution européenne, qui donnera à notre gouvernement un appui lors les négociations difficiles qui se rouvriront dans les mois prochains à Bruxelles. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à excuser ma collègue Cécile Cukierman qui devait prendre la parole aujourd'hui, mais qui est retenue dans la Loire. Faire mieux avec toujours moins de moyens » : monsieur le ministre, si je devais résumer en une seule phrase la direction prise pour l'avenir de la PAC, ce serait celle-là.

Ajoutons à cela une baisse du budget et vous voyez combien l'avenir de cette PAC, pourtant politique européenne historique, est sombre. Alors, oui, les objectifs annoncés par la Commission européenne sont louables sans faire de liste exhaustive, nous pouvons nous féliciter de la volonté annoncée d'assurer un revenu équitable aux agriculteurs, de rééquilibrer les pouvoirs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, ou encore d'agir contre le changement climatique. Mais soyons sérieux comment réaliser tout cela avec un budget amputé de près de 16 % et, surtout, sans instrument de régulation ? À l'heure où la Commission européenne fait des annonces vertueuses, l'Union multiplie les accords de libre-échange- seize sur la table -, alors que, comme nous le disons depuis longtemps, il est temps d'en finir avec ce modèle économique de libre-échange. Celui-ci nuit aux agriculteurs comme aux citoyens et, surtout, les conséquences environnementales sont désastreuses. Pourtant les États généraux de l'alimentation ont montré que l'on a impérativement besoin de construire un nouveau modèle fondé sur la recherche de la qualité et sur la relocalisation de productions créatrices d'emploi. Le CETA va exactement dans le sens opposé des objectifs annoncés ... comme une certaine loi Égalim. Alors, monsieur le ministre, est-ce un discours de façade ou l'expression Je laisse à chacun le soin de se faire son avis. De plus, la Commission européenne a même précisé que « l'aide aux agriculteurs ne doit pas avoir ou peu d'incidences sur les échanges commerciaux pour que l'Union puisse respecter ses obligations [ ...] dans l'accord de l'Organisation mondiale du commerce ». Elle fait donc fi de la question de la rémunération des agriculteurs, de la régulation du fonctionnement des marchés et de la volatilité des cours des produits agricoles.

ne définit pas de politique européenne en termes d'échanges avec le reste du monde : à défaut de définir des tarifs douaniers ou des règles d'importation des produits agricoles venant d'autres zones du monde, cette PAC s'inscrit dans un marché mondialisé et dérégulé. Dès lors, je ne peux que me féliciter de la qualité du rapport conjoint de la commission des affaires européennes et de la commission des affaires économiques, qui ne se sont pas trompées. Oui, mes chers collègues, la réforme qui se profile sera un coup fatal porté à notre modèle agricole. Pour la première fois, la PAC va peu à peu être dissoute au profit des politiques agricoles nationales, variant d'un pays à l'autre, tout comme va l'être l'idéal européen, qui était de construire une destinée agricole commune. Cet abandon se reflète d'ailleurs dans la position de la Commission européenne tout comme dans celle du gouvernement français. Lors des négociations, monsieur le ministre, vous avez mis en avant la nécessité de préserver un budget stable, ce qui est certes impératif, mais vous semblez avoir oublié que les modalités de gestion de la PAC sont tout aussi importantes importantes et déterminantes. Au travers d'un nouveau mode de gestion censé être moins bureaucratique, c'est l'approche uniforme, jusqu'ici en vigueur, qui est remise en cause, remplacée par des plans stratégiques élaborés par les États membres, puis validés par la Commission. Chaque pays pourra ainsi définir des objectifs en compétition avec ceux de ses voisins, ce qui introduira de fait un risque de dumping puisque les règles environnementales, mais aussi sociales, peuvent être adaptées. Dans cette nouvelle PAC, seuls les grandes firmes agroalimentaires et les grands acteurs de la distribution seront en mesure d'avoir des projets à dimension européenne, à grand renfort de rachats et de fusions-acquisitions. À l'opposé, nous prônons une PAC à l'échelle européenne, afin de permettre une transition vers l'agriculture paysanne et le maintien de paysans nombreux sur tous les territoires. Face au défi climatique et alimentaire, c'est d'une PAC ambitieuse et rénovée que les Européens ont besoin, et cela implique la reconnaissance d'une exception agricole, l'exclusion du secteur agricole des accords de libre-échange et l'indispensable besoin d'une coopération fondée sur des objectifs partagés. Nous devons sortir la PAC de cette politique productiviste mortifère. À l'inverse, les Français et les Européens dans leur ensemble veulent une agriculture favorisant les circuits courts, permettant une meilleure traçabilité des produits et favorisant de nouvelles formes de distribution. de nouvelles formes de distribution. Ce qu'ils veulent surtout, c'est une redirection des aides vers les exploitations paysannes en faveur de la transition écologique et une sortie du glyphosate et des substances nocives pour la santé. Pour conclure, les Européens veulent non pas d'une PAC au rabais, mais d'une PAC en faveur de l'emploi paysan et d'une transition vers l'agriculture paysanne,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette nouvelle proposition de résolution européenne sur la réforme de la PAC reprend quelques-uns des grands principes formulés dans les deux textes que le Sénat avait successivement adoptés en 2017 et 2018, et que nous avions pour la plupart approuvés. Pourquoi renouveler aujourd'hui une attention soutenue sur cette question ? Parce que nous mesurons, au Sénat, combien il est fondamental d'encourager une agriculture performante et durable à l'échelle européenne et de garantir l'avenir des exploitations dans nos territoires. Est-il utile de rappeler tous les enjeux que recouvre l'agriculture ? J'ai déjà eu l'occasion de les énumérer : indépendance alimentaire, qualité des produits agricoles, santé publique, emplois non délocalisables, exigences environnementales et aménagement du territoire, sans oublier une réponse aux mutations sociétales et aux attentes des consommateurs. Cela invite à poursuivre avec détermination notre travail d'alerte face aux difficultés, comme la volatilité des prix et les crises sanitaires et climatiques : rares sont les secteurs économiques qui cumulent autant d'aléas. Ce contexte génère un mal-être qui pousse trop souvent nos paysans au geste fatal : un agriculteur se suicide tous les deux jours. Je ne cesserai de le répéter tant ce chiffre, qui ne fait pas l'actualité, Pourtant, la filière ne ménage pas sa peine, consciente depuis bien longtemps des mutations. De PAC en PAC, les paysans jouent le jeu de l'adaptation. Quand il a fallu produire plus dans les années 1960, ils l'ont fait. Quand on leur a demandé de produire moins avec les quotas, ils l'ont fait aussi. Aujourd'hui, on leur demande de produire mieux. Beaucoup le font déjà, et les autres attendent tout simplement qu'on leur en donne les moyens. La PAC pour 2021 à 2027 va-t-elle dans le bon sens ? Les propositions européennes, publiées par la Commission le 1 juin 2018, donnent-elles les clefs pour une agriculture à la fois compétitive, rémunératrice et respectueuse de l'environnement ?

seulement 3 % des 700 millions d'euros dédiés au programme Leader ont été consommés. C'est un gâchis 100 % français, car nous avons un gros problème qui se résume en une simple phrase : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Les territoires ruraux font les frais d'une complexification, mais aussi d'un transfert de gestion de ces dossiers aux régions, alors que celles-ci n'y avaient pas été préparées. À un an de la perte de ce budget, la solution est urgente : simplifier les modalités d'instruction. Sur la prochaine PAC, tout a été dit. On ne peut se satisfaire d'une baisse de 15 % des crédits par rapport au budget 2014-2020. Sans méconnaître les nouvelles priorités de l'Union européenne, l'agriculture ne doit pas devenir la variable d'ajustement. Cette diminution est à contre-courant de ce que font les grands pays, comme les États-Unis, la Chine et le Brésil, qui renforcent au contraire les moyens qu'ils consacrent à l'agriculture, bien conscients de son rôle stratégique, sans oublier les logiques d'accaparement des terres dans lesquelles certains s'engagent aussi. Se profile le défi alimentaire global d'un monde à 9 milliards d'individus d'ici à 2050, auquel l'Union européenne devra prendre toute sa part. Il faut nous y préparer dès aujourd'hui. Le métier d'agriculteur est un métier d'avenir. La question des moyens de la PAC est aussi pour chacun des États membres celle du niveau des aides que l'on peut apporter à nos agriculteurs à l'échelon local pour soutenir leurs revenus, ainsi que les transitions qu'ils doivent opérer sur leurs exploitations. Dans le cadre de la loi Égalim, nous avons beaucoup discuté de la question des revenus, car il n'est plus admissible que les agriculteurs vivent à peine, ou plus du tout, de leur travail et se retrouvent victimes de la guerre des prix de la grande distribution. Sur ce point, j'en profite pour saluer les avancées du projet de directive sur les pratiques commerciales déloyales, qui accentuera ce que l'on a pu déjà faire au niveau national. Pour revenir à la PAC, je note avec satisfaction un meilleur ciblage des aides au sein de la nouvelle architecture des paiements. En parallèle, il faut mettre en place un système très opérant de gestion des crises, ce qui implique de reconquérir les esprits au niveau européen pour que le mot « régulation » ne soit pas tabou. On se souvient de l'attentisme des institutions européennes lors de la crise du lait en 2015. Par ailleurs, la PAC n'a de sens que si elle garantit aussi pour ses agriculteurs un cadre intra-européen de concurrence loyale. À cet égard, la proposition de résolution insiste sur le principal écueil du nouveau mode de mise en oeuvre de la PAC, qui instaure davantage de subsidiarité. Mais la Commission est-elle prête à revoir sa copie pour éviter que ne s'instaure un dumping social ou normatif, lequel serait notamment défavorable aux exploitants qui s'engagent dans la transition agroécologique ?

La proposition de résolution en faveur de la création de paiements pour services environnementaux va dans ce sens. Je l'ai cosignée avec mes collègues Franck Montaugé et Jean-Claude Tissot, mais cette proposition est également soutenue par Joël Labbé, qui a d'ailleurs organisé un colloque au Sénat pour la mettre Ce serait un juste retour des choses, pour tout ce qu'apportent à la collectivité les milliers de femmes et d'hommes qui s'investissent au quotidien dans leurs exploitations. À l'heure de l'agribashing, au lieu de stigmatiser nos paysans, il faut soutenir ceux qui ont opté pour des modes de production vertueux. Les conclusions du rapport 2019 de l'IPBES sur la perte de la biodiversité nous obligent à une responsabilité commune, notamment dans le cadre d'une politique européenne d'agriculture durable que nous devons coconstruire avec tous les États membres.

obligés de tronçonner leurs arbres face la commercialisation d'oranges provenant d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Nous sommes tous concernés et nous devrions être tous solidaires face à l'iniquité des charges sociales et des cahiers des charges concernant les modes de production, en adoptant une réelle politique commune qui lisse déjà en interne les obligations de chacun. Enfin, je pense vraiment qu'il faut exclure les produits alimentaires des accords de libre-échange, car on ne peut absolument pas garantir une transparence sur ces produits à l'heure actuelle. En attendant ces avancées, le RDSE approuvera la proposition de résolution européenne sur la prochaine réforme de la PAC, que nous souhaitons, d'un mot, plus ambitieuse. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour la France, première puissance agricole de l'Union européenne, la PAC constitue un enjeu majeur : un enjeu alimentaire, un enjeu économique, un enjeu d'aménagement du territoire. nous examinons aujourd'hui une troisième proposition de résolution, les deux premières ayant été peu ou pas entendues. À l'heure où l'Union européenne doit s'affirmer face aux pressions américaines ou asiatiques, il nous apparaît essentiel de ne pas manquer le rendez-vous de la PAC de 2020. Cette réforme doit être à la hauteur du nouvel ordre mondial qui se dessine. Pour s'imposer, l'Union européenne doit s'appuyer sur ce qui constitue le socle de sa cohésion, la politique agricole commune, et affirmer très clairement une vision stratégique pour l'agriculture de demain. Comment alors admettre une PAC qui s'orienterait vers une diminution de plus de 15 % des aides directes, bien au-delà des 13 milliards d'euros induits par le Brexit et qui se traduirait par des baisses importantes de revenus des agriculteurs ? Quand nous savons qu'un tiers des agriculteurs français vivent avec moins de 350 euros par mois, ces perspectives ne sont pas acceptables, d'autant qu'elles s'inscrivent- nous le savons -dans une mondialisation et une dérégulation grandissantes des marchés, qui font peu de cas des standards européens et d'une concurrence loyale. Monsieur le ministre, quelles sont les chances de survie de notre modèle agricole familial et extensif dans un tel contexte ? Avec, qui plus est, un risque de renationalisation des politiques et le retour en force des stratégies du moins-disant, de dumping social et environnemental, pour conquérir les marchés du voisin. On s'interroge : où est la vision communautaire ? Soyons donc plus cohérents ! Nous avons voté, il y a quelques mois, une loi Égalim, qui préconise la contractualisation, le regroupement en organisations de producteurs, une montée en gamme, l'inversion de la construction du prix et une meilleure répartition de la valeur entre producteur, transformateur et distributeur. Pour mettre en place cette loi et être cohérents, il nous faut une PAC qui protège et qui permette d'agir pour une meilleure reconnaissance et une plus juste rémunération du producteur, lui permettant de vivre dignement de son métier, mais aussi-vous l'avez dit, monsieur le ministre -d'investir, d'innover et de gagner en compétitivité agricole. Les citoyens, les élus, les consommateurs veulent une PAC forte et ambitieuse, mais également réaliste, et non une PAC de repli face aux puissances agricoles conquérantes, américaine, asiatiques ou russe, celles-là mêmes qui semblent avoir bien saisi toute la dimension hégémonique de l'enjeu agricole dans les prochaines décennies et investissent massivement. Ils veulent une PAC qui s'adapte sans ignorer les pratiques protectionnistes grandissantes de ces mêmes acteurs, lesquels viennent conquérir les marchés européens mais protègent les leurs. Nous concluons acteurs des accords de libre-échange portant sur nos filières les plus vulnérables, parce que les plus exigeantes en qualité- je pense notamment au piège dans lequel nous poussons nos producteurs de viande et ce sans respecter l'article 44 de la loi Égalim, qui interdit la vente de produits alimentaires ne respectant pas les normes de production ou de traçabilité européennes. Avec cette nouvelle PAC, cela a été dit, c'est ni plus ni moins la subsistance du modèle d'agriculture français, mais aussi européen, familial, extensif, de qualité et de proximité, présent sur l'ensemble de nos territoires, nourrissant les populations et exportant dans le monde entier, qui est en jeu. Ce modèle crée des emplois et aménage le territoire. C'est la raison pour laquelle le Sénat réaffirme une fois de plus, en cette période cruciale, que le rendez-vous de la réforme de la PAC ne doit pas être manqué. Comme ses prédécesseurs l'ont fait avec succès, le Président de la République doit lui-même peser dans les négociations à venir et tracer la voie de l'agriculture européenne du XXI siècle, compétitive et responsable.

la qualité des productions, la santé des consommateurs et le respect de l'environnement deviennent les maîtres mots. Pour le groupe Union Centriste, qui apporte son total soutien à cette résolution, c'est ainsi que la France apportera sa contribution à une Europe agricole plus juste et plus responsable, une Europe forte qui relève les défis du XXI siècle, faisant écho aux attentes clairement exprimées par les jeunes générations. Mes chers

soit le plus haut niveau depuis 2010, c'est-à-dire 15 % de plus qu'en 2018. Monsieur le Premier ministre, vous menez, avec le Gouvernement et la majorité, une politique active en faveur de l'emploi. L'OCDE souligne souligne les effets positifs des lois et des mesures qui ont été prises, et elle nous encourage à poursuivre dans cette voie, tout en prenant soin de tous les problèmes sociaux qui se posent à côté et que nous n'ignorons pas. une trop grande partie de notre jeunesse, de nos seniors et de certains de nos territoires restent exclus du monde du travail. Doit-on donc penser qu'il s'agit d'une fatalité, malgré les efforts entrepris pour redonner au travail la place qu'il mérite ? ? Hier, à Matignon, monsieur le Premier ministre, devant les partenaires sociaux et les élus locaux, vous avez rappelé votre objectif : une mobilisation totale pour l'emploi et des solutions concrètes apportées à des problèmes concrets. Il y va de la responsabilité de chacun d'entre nous. Il serait temps ! Sans doute, mon cher collègue, mais il y a encore, aujourd'hui, des apprentis qui, malgré les lois, ne trouvent pas les solutions dont ils ont besoin. Nous devons agir dans la concertation, pour lever les freins quotidiens à l'embauche, au déplacement, à la formation et multiplier les emplois liés à la transition écologique. À ce titre, la journée d'hier a posé les bases d'une démarche. Pouvez-vous nous dire, monsieur le Premier ministre, en précisant le cadre, la méthode, le calendrier et les responsables, comment seront mises en place ces actions nécessaires et attendues de tous ? La parole

président Patriat. Elle va me permettre d'indiquer le sens et le fonctionnement de la démarche engagée hier à Matignon, à l'occasion du lancement de la mobilisation nationale et territoriale pour l'emploi et les transitions.

d'un seul- une seule collectivité, l'État seul, un syndicat ou les seules entreprises -et que, pour lever les freins au retour à l'emploi, pour favoriser encore plus le recours à l'apprentissage, pour mettre en oeuvre les instruments de la transition écologique au quotidien, il fallait, indépendamment de la définition de nouveaux instruments ou de la sollicitation de nouveaux budgets, mobiliser les acteurs, afin de trouver des solutions concrètes. Nous avions identifié cinq thèmes, cinq sujets, sur lesquels nous pouvons nous réjouir d'un certain nombre de nouvelles. Le premier, c'est l'apprentissage. Vous avez raison,

un certain nombre de questions pratiques continuent de constituer des freins au développement de l'apprentissage. Comment faire en sorte que toute personne voulant obtenir un contrat d'apprentissage trouve une entreprise pour l'accueillir ?

On ne peut répondre à ces questions qu'en rassemblant autour de la table l'ensemble des partenaires intéressés par leur résolution. Je pense ainsi aux collectivités territoriales, aux associations aux associations environnementales et sociales, aux organisations syndicales et patronales ; en outre, pour la réunion que j'ai organisée hier à Matignon, j'avais demandé à un représentant du Sénat- ce fut le sénateur Dallier -et à un représentant de l'Assemblée nationale d'être présents, afin que l'ensemble des institutions et des et des partenaires puisse travailler concrètement à la définition de ces solutions. Nous avions identifié, je l'ai dit, cinq sujets ; il est apparu opportun, lors de la discussion, d'en ajouter un sixième, celui de la rénovation thermique des bâtiments. les organisations syndicales et les associations environnementales nous ont dit que, malgré l'existence de budgets, d'instruments et de compétences dédiés, c'était encore trop compliqué, qu'il y avait encore trop de freins pour déclencher les décisions de rénovation thermique des bâtiments. Il nous faut donc trouver des solutions concrètes. Nous sommes convenus d'une méthode Nous sommes convenus d'une méthode : les préfets de région et les présidents de conseil régional organiseront, conjointement, des mobilisations territoriales avec l'ensemble des partenaires.

Notre objectif est simple, mesdames, messieurs les sénateurs : faire en sorte que les questions concrètes trouvent des réponses concrètes. En juin, une fois le travail fait en région, il sera possible de déterminer

les directeurs départementaux des finances publiques ont reçu, en décembre 2018, une note interne intitulée « Bâtir un nouveau réseau ». Cette note prévoit le démantèlement du réseau de proximité des finances publiques, avec, notamment, la suppression des trésoreries et le regroupement des services des impôts des particuliers et des services des impôts des entreprises d'ici à 2022. Ainsi, dans le département dont je suis élue, le Cantal, l'application de ce projet pourrait avoir des conséquences très importantes, avec la fermeture de treize trésoreries, de deux services des impôts des particuliers et de deux services des impôts des entreprises. Ces suppressions aggraveraient évidemment la fracture territoriale qui pénalise déjà très lourdement de nombreux territoires ruraux, dont la population, en moyenne plus âgée qu'ailleurs, rencontre de réelles difficultés dans l'utilisation de l'outil numérique. Ne l'oubliez pas, la couverture numérique du territoire n'est pas encore achevée, ce qui contribue à pérenniser les inégalités territoriales La présence physique de personnel compétent y est donc indispensable, au nom de la conception du service public à laquelle nous sommes attachés. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner plus d'informations sur la suppression envisagée des services de proximité des finances publiques et nous indiquer comment vous comptez les remplacer

Les 2 500 trésoreries et les 110 000 agents des finances publiques seront au plus près des territoires ; moins de personnes à Paris, plus de personnes dans le Cantal, voilà, pour résumer, la politique du Gouvernement. La parole est

Le droit constitutionnel de manifester dans le respect est essentiel dans une démocratie. Sans casser ! Pourtant, il a été bafoué à Paris, le 1 mai. Les victimes des interventions violentes et répétées dues, pour l'essentiel, aux forces de l'ordre furent les dizaines de milliers de manifestants réunis ce jour, et non les Black Blocs, dont nous condamnons tous les actes. Cette violence fut déclenchée dès le départ de la manifestation, et- fait inédit -les cortèges syndicaux furent la cible de tirs de grenades et se retrouvèrent noyés dans un nuage de gaz lacrymogène. J'y étais, monsieur le Premier ministre, et j'ai été le témoin de cette agression irresponsable contre des manifestants. À la télévision et sur Twitter, M. Castaner a d'abord évoqué une « attaque » contre l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et a même affirmé que nos « forces de l'ordre [étaient] intervenues pour sauver le service de réanimation ». Or les faits et rien que les faits démontrent le contraire. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas employé les mêmes termes, mais vous avez indiqué, le lendemain, que le « fait d'entrer dans un hôpital alors qu'on est en train de manifester est idiot et, au fond, scandaleux. » Je ne qualifierai pas ici l'intelligence des propos de M. Castaner, mais pouvez-vous enfin reconnaître

Où est la République de la responsabilité, souvent convoquée par le Président de la République ? Je le dis avec force, tout cela n'est pas qu'une question de sémantique. La crédibilité du ministre de l'intérieur, qui a manipulé l'opinion, est aujourd'hui entachée, et il devrait, pour le moins, être entendu par les commissions des lois du Parlement.

est organisée, dans le droit français, comme toutes les libertés publiques, et, comme toutes les libertés publiques, elle s'exprime dans le respect du droit. Bien sûr ! J'observe que, depuis le début de ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement des « gilets jaunes des gens qui se réclament de la liberté de manifester prennent un soin infini à ne pas respecter les règles posées par les parlementaires et par la jurisprudence sur le droit de manifester.

non pas du tout de conjuguer leurs efforts pour cette commémoration et pour cette manifestation, mais bien de casser, de provoquer, de profiter de la manifestation pour faire bien autre chose. Nous en

C'est ce que nous avons fait, ... Non ! ... en donnant des consignes et en organisant les choses de telle façon que les Black Blocs, comme vous les appelez à juste titre, ne puissent pas venir se mélanger, ne puissent pas priver de leur droit ceux qui veulent manifester dans le respect des règles. C'est évidemment un exercice difficile

je considère que, de ce point de vue, la journée du 1 mai dernier a été remarquablement tenue. En effet, le ministre de l'intérieur, le préfet de police, l'ensemble de la chaîne de ceux qui sont intervenus en matière d'ordre public ont permis d'éviter les débordements qui étaient pourtant annoncés,

une intrusion et, à l'évidence, un certain nombre de gens qui étaient présents sur les lieux ont d'abord dit que cette intrusion violente leur avait leur avait donné le sentiment que le fonctionnement normal du service de réanimation- lequel est évidemment sensible, je pense que vous en conviendrez -serait mis en cause ; cela aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Compte tenu de ces informations, le ministre de l'intérieur a fait une déclaration. Très rapidement, le lendemain, il a indiqué que, compte tenu ce qu'il savait, il avait utilisé une expression qui n'était pas adaptée.

Le corriger, en assumant d'avoir utilisé un terme qui n'était pas adapté et en revenant à un terme qui l'est parfaitement, fait honneur à celui qui le fait, c'est une bonne chose et cela me semble à la hauteur de ce que doit faire un responsable politique. Je veux donc, à cette occasion, redire toute ma confiance en M. le ministre de l'intérieur. La parole

avons entendu vos explications et nous partageons la condamnation de ceux qui utilisent les manifestations pour casser et dévoyer les revendications légitimes de ceux qui s'expriment par ce biais. rien ne peut justifier qu'un ministre de l'intérieur, qui est là pour apaiser et permettre la concorde, jette de l'huile sur le feu en proférant un mensonge massif. Rien ne peut justifier qu'on utilise des techniques de nasse, dont des manifestants légitimes, travailleurs, femmes, enfants, ne peuvent s'échapper.

la liberté de manifester malgré la présence de casseurs ? Je le dis solennellement ici : ma génération n'oubliera jamais Malik Oussekine et la façon dont il a été tué, à quelques dizaines de mètres d'ici, en se réfugiant dans une cage d'escalier.

heures, nous avons ouvert le chemin, et les 18 000 premières personnes n'ont pas bougé ; alors, nous avons mis en place une force intermédiaire entre la tête du cortège et le cortège de la CGT et des autres partenaires sociaux, pour les faire avancer.

! » Monsieur le sénateur, vous me faites un reproche, celui d'avoir choisi un mot, « attaque », à partir des témoignages qui venaient de m'être livrés par le personnel hospitalier. Au vu des éléments apparus le lendemain, j'ai corrigé ce mot, et je l'ai fait sans aucun état d'âme,

Alors que l'homme en est le principal responsable, sommes-nous à la hauteur pour arrêter ce désastre et en protéger les générations qui viennent ? La biodiversité n'est pas un catalogue d'espèces ni une obsession d'écolo à la mode ; ce n'est pas un sujet d'actualité ni un argument de campagne ; c'est un « miracle » qui a nécessité quelques milliards et plusieurs centaines de millions d'années d'évolution.

Les dossiers des Dreal et des DDT sont remplis de demandes d'artificialisation des sols, qui sont la plupart du temps approuvées, toujours pour de bonnes raisons ... Ainsi, tous les cinq ans, la surface agricole utile équivalente à un département disparaît Quand arrêterons-nous définitivement de morceler nos campagnes, de polluer nos rivières, de détruire les myriades d'étangs et autres zones humides qui sont la richesse de notre pays ? s'accumulent sur les étagères des ministères des rapports sur l'extinction de la biodiversité et sur les solutions pour y mettre fin. Pour nous rassurer, depuis des années, tous les gouvernements successifs s'étourdissent de mots, de réunions, de colloques, de plans d'action. Monsieur le ministre d'État, le Parlement a les mains liées ; la Constitution confie au Gouvernement la charge de l'urgence et de l'ordre du jour prioritaire. C'est aussi le Gouvernement qui a les clefs de Bercy. Pouvez-vous donc nous annoncer le calendrier de la mise en oeuvre des dispositions destinées à arrêter la perte irréversible de ces millions d'insectes, d'oiseaux, de mammifères qui peuplent notre planète ? La parole

beaucoup de gens ridiculisaient un tel engagement : « À quoi bon s'intéresser aux petites fleurs et aux petits oiseaux ? Il y a bien d'autres sujets beaucoup plus importants. Or, aujourd'hui, des scientifiques du monde entier ont fait un rapport précis sur l'état de la biodiversité ; cela passe, en effet, par la mesure des petites fleurs et des petits oiseaux, chez nous, en France, comme partout dans le monde. d'être un ministre nommé par un Président de la République qui a reçu ces scientifiques. C'est la première fois qu'un Président de la République fait de la biodiversité un enjeu dans la politique internationale, dans la diplomatie française, de même niveau que le climat. Par ailleurs, demande au Gouvernement d'agir, ici et maintenant, dans sa politique pour la biodiversité. Je veux vous donner deux exemples pour garder espoir, car vous m'avez semblé céder un peu au fatalisme ; pour ma part, je ne céderai jamais au fatalisme sur ce sujet. Dans les années 1970

Parce que nous avons su prendre des mesures de prévention, de lutte contre les problèmes de pollution, à la racine. En matière d'eau, il s'agit de la lutte contre les pollutions industrielles et de l'amélioration du traitement des eaux usées,

La parole est à M. Philippe Bas, pour le groupe Les Républicains.

mai dernier, plusieurs dizaines de manifestants ont pénétré, certains par effraction, dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour échapper aux gaz lacrymogènes. Cette irruption dans un lieu de soins était de nature à susciter une légitime émotion. Heureusement, aucune agression ne semble avoir été commise, et les manifestants n'ont apparemment pas pénétré dans les bâtiments. Je veux saluer ici le sang-froid, le calme et le formidable professionnalisme dont ont fait preuve les personnels de santé pour maintenir les patients à l'abri de cette agitation qui a fait peur. Las, on ne peut dire que le Gouvernement ait fait preuve du même sang-froid si l'on en juge par ses déclarations On a attaqué un hôpital », « on a agressé son personnel soignant », « c'est une intrusion violente », avez-vous dit successivement, monsieur le ministre. « C'est un acte scandaleux avez-vous ajouté, monsieur le Premier ministre. « C'est une exaction inqualifiable et indigne », a déclaré la ministre de la santé. Quant au président de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l'ancien ministre Le Guen, il a ajouté : « C'est un acte de pure barbarie. » Alors, monsieur le ministre, sur quels faits le Gouvernement s'est-il fondé pour donner l'alarme aux Français sur des violences qui n'ont pas eu lieu ?

les responsables hospitaliers qui m'ont accueilli m'ont fait part de leur émotion. C'est sur la base de leur émotion, filmée par les chaînes d'information, que je me suis prononcé. C'est sur la base de cette émotion extrêmement forte que j'ai dénoncé ces faits. Monsieur Bas, jamais, je crois, dans l'histoire d'une manifestation,

Madame la ministre de la cohésion des territoires, lors de sa conférence de presse du 25 avril dernier, le Président de la République a annoncé une disposition en faveur des milieux rural et périurbain, le déploiement de maisons de services au public sous la nouvelle appellation « France service ». Notre pays compte déjà plus de 1 300 maisons de services au public qui permettent non seulement de pallier la fermeture de services publics, mais aussi la fracture numérique dans certains territoires. Mises à disposition par les collectivités territoriales, aidées par l'État et par différents organismes publics ou privés, ces maisons de services au public sont, sans aucun doute, un gage d'attractivité du territoire lorsque leur fonctionnement et leur organisation sont bien assurés. Le Président de la République a annoncé leur déploiement à raison d'un France service par canton. Je m'interroge sur cette intention. En effet, le dispositif mis en place sur l'initiative des communes et des EPCI avait pour objectif de constituer un bon maillage territorial. Il n'est pas rare de compter deux ou trois maisons de services au public dans certains cantons ruraux, en raison de leur étendue ou, tout simplement, de l'existence de bassins de vie dépassant les limites administratives du canton. Ne pensez-vous pas, madame la ministre, que le principe d'un seul France service par canton aboutisse à un affaiblissement du dispositif existant ? Toutefois, la question essentielle me semble être celle du financement : depuis quelques mois, les projets en cours sont gelés, faute de crédits. Pouvez-vous nous indiquer les dispositions financières qui permettront de mettre en oeuvre ces engagements du Président de la République ? Enfin, compte tenu de la situation particulière des territoires ultramarins,

constituent le prolongement naturel des maisons de services au public, souvent encore trop peu connues de nos concitoyens et qui correspondent à un réel besoin de proximité, largement exprimé lors du grand débat. grand débat. Il existe aujourd'hui 1 340 maisons de services au public sur l'ensemble du territoire. Le Premier ministre a annoncé la création de 500 nouvelles maisons. Au regard du maillage actuel,

des faits « cruels » et la nécessité de changer de modèle économique de production. Il n'est pas le premier à trouver les mots. Tout le monde se rappelle l'orfèvre en la matière que fut Jacques Chirac, lors du sommet de la Terre, à Johannesburg. à Johannesburg. À l'inverse de ses prédécesseurs, qui ont finalement beaucoup laissé brûler la maison, Emmanuel Macron sera-t-il le premier à définir et appliquer des politiques publiques à la hauteur de ces défis redoutables ? La crédibilité de la réponse passera par des actes, rien que par des actes, et par de vrais investissements. À l'heure où, mû par une légitime émotion, notre pays se mobilise pour reconstruire une cathédrale au coeur de son histoire, l'État peut-il laisser se perdre des pans entiers de son patrimoine naturel ? 120 espèces endémiques sont en danger d'extinction en France, notamment dans les territoires ultramarins, où beaucoup de ces espèces se portent bien plus mal que le bouquetin dans les Alpes. Nous avons voté, dans la loi Biodiversité, et j'ai eu l'honneur de porter cet amendement, un article disposant que toutes ces 120 espèces devraient, d'ici au 1 janvier 2020,

Vous posez une question précise sur les espèces endémiques en danger, qui doivent faire l'objet, comme vous l'avez souligné, depuis la loi Biodiversité de 2016, de plans de protection, dits plans nationaux d'action, ou PNA. Nous avons lancé 65 PNA, dont 16

objectif, et il est important.

Les Républicains. Ma question s'adresse à Mme la ministre des solidarités et de la santé. Madame la ministre, lors de l'examen du PLFSS pour 2019, votre collègue chargé du budget annonçait fièrement que le bon vieux trou de la sécurité sociale, qui aggrave les déficits publics depuis 2002, allait être rebouché. Et cela, dès 2019, disait-il, avant le retour à l'équilibre promis par le Premier ministre dans son discours de politique générale. Je vous ai bien écoutée

à la fin de l'année, un déficit de 3,6 milliards d'euros. C'est ce qu'annonce le Haut Conseil du financement de la protection sociale, dans son rapport du mois de mars. Il y précise même qu'aucun équilibre n'est envisageable avant la fin du quinquennat. Les promesses d'un petit excédent de 600 millions d'euros se sont envolées, le discours de la fin de l'année a été happé par la réalité. Comment, madame la ministre, pouvez-vous expliquer et justifier un tel décalage entre les prévisions présentées comme la preuve incontestable de la bonne gestion du Gouvernement et la réalité des chiffres de la fin de l'année 2019 ? Quels objectifs se fixe désormais le Gouvernement en termes de réduction du déficit de la sécurité sociale ? comment allez-vous, en l'absence d'excédents, financer les nouveaux moyens confiés à la CADES, qui n'avaient été déclarés conformes à la Constitution qu'en raison des excédents prévisionnels du budget de la sécurité sociale

l'anticipation, en janvier 2019, de l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires représente un manque de 1,3 milliard d'euros

Le Gouvernement a fait le choix d'une communication sur le maintien de l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Dire la vérité aux Français sur la nécessité de prolonger l'effort entrepris par les précédentes réformes me semble être de nature à créer la confiance.

Cette rencontre avait pour objet de célébrer la personnalité universelle de Léonard de Vinci, mort voilà cinq cents ans. Cet évènement symbolique rappelait l'amitié franco-italienne, quelque peu mise à mal, et surtout préfigurait, en en donnant le coup d'envoi, les festivités des cinq cents ans de la Renaissance en Val de Loire. Tout portait donc à s'attendre à un moment festif pour la population ... Las, une tornade sécuritaire s'est abattue sur la ville. Je ne résiste pas à l'envie de vous détailler les consignes passées aux habitants

Cette ville touristique de 13 000 habitants, très active, accueillant près de 1 million de visiteurs par an, s'est trouvée bouclée et désertée. Une ville fantôme vidée de toute vie, un véritable désert, commentent les habitants bloqués chez eux. Tous les commerces ont leur rideau baissé. Une ambiance aussi impressionnante que ridicule ... Ô combien ! On peut rétorquer qu'une menace terroriste est toujours présente. Ressort alors l'image de la visite du général de Gaulle, en 1959, émergeant d'une marée humaine en liesse, au pied du château. Vu de Paris, vu de Rome, cette ville « sous cloche », comme le titrait le journal local, marquait peut-être un signe fort de l'amitié franco-italienne, mais, vu d'Amboise, c'était la sidération, l'image d'une ville parfaitement vide. Il faut conclure ! Il y a donc des questions à se poser sur les rapports d'un Président avec le peuple et de ce pouvoir avec la nation. Le traitement de la sécurité Le traitement de la sécurité par le vide est-il vraiment nécessaire ? S'agit-il, là aussi, d'une nouvelle doctrine sécuritaire pour les déplacements présidentiels ?

En novembre 2018, le Président de la République s'était prononcé favorablement pour la mise en place d'une taxe flottante « anti-pic » pour lutter contre l'augmentation exponentielle du prix des carburants. Aucune suite n'y a été donnée ... Or c'est bien cette augmentation des prix de l'essence qui avait déclenché le mouvement social des « gilets jaunes », à l'automne dernier- mouvement qui, à ce jour, continue de mobiliser. Devant la poursuite de cette hausse des prix du baril, et malgré le gel de la taxe carbone, vous avez exprimé, mardi dernier, votre refus de recourir à une taxe flottante sur les carburants. Initiée sous le gouvernement de Lionel Jospin et instaurée encore à l'été 2012, par voie d'arrêté, pour une période de trois mois, cette taxe permet de réduire instantanément le prix à la pompe de 3 ou 4 centimes.

J'ai évoqué la taxe flottante, mais d'autres mesures pourraient être actionnées en direction des marges des distributeurs, lesquels, me semble-t-il, ne traversent pas de crise majeure, bien au contraire. Je pense surtout aux grands groupes pétroliers, dont les bénéfices sont en forte hausse, pour ne pas dire explosifs, ces dernières années. Eux aussi devraient pouvoir contribuer à la transition énergétique, ce qui allégerait d'autant la fiscalité pesant sur les ménages. L'effort fiscal doit incontestablement être mieux réparti. Ma question est donc très simple : quelles solutions, à court terme, le Gouvernement est-il en mesure de proposer pour épargner aux Français une nouvelle ponction excessive sur leur pouvoir d'achat en raison de l'augmentation du prix du baril ?

Vendredi dernier, j'ai eu le privilège de suivre, pendant plus de huit heures, un équipage de la BST nord, puis de la BAC centre de Marseille. J'ai pu observer de près leur travail au coeur des « supermarshits », ces cités où le trafic de drogue peut rapporter jusqu'à 60 000 euros par jour et où les racailles jouent de la Kalach en plein après-midi. Ces rues de Marseille où, à la nuit tombée, il ne fait vraiment pas bon être une femme seule, être juif ou homosexuel, ou tout simplement être « de souche ». Dans les deux cas, j'ai constaté que ces policiers n'ont qu'un objectif : garantir à nos compatriotes la première des libertés qu'est la sécurité, et cela souvent au péril de leur vie. J'ai posté sur mes réseaux sociaux un bref compte rendu de cette expérience. Quelle ne fut pas ma mauvaise surprise de lire de trop nombreux commentaires d'hostilité envers les forces de l'ordre, motivés par les blessures dont ont été victimes certains « gilets jaunes ». Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment un tel fossé a-t-il pu se creuser entre la police et une partie de la population, alors que le soutien populaire était unanime depuis les attaques, réelles celles-là, des terroristes islamistes qui ont fait plusieurs victimes, je le rappelle, parmi les forces de l'ordre ? Ce fossé, pour ne pas dire ce projet, a débuté en novembre 2018, quand vous avez appliqué avec zèle la stratégie établie par Emmanuel Macron du pourrissement du mouvement légitime, et au départ pacifique, des « gilets jaunes « gilets jaunes ». Vous avez laissé s'y infiltrer la violence venue de groupes d'anarchistes et d'extrême gauche que vous refusez toujours de dissoudre. Par calcul politique et électoral, vous avez volontairement dressé les Français les uns contre les autres, quitte à sacrifier l'image de la police, n'hésitant pas à « bluffer », comme on dit chez vous, autrement dit à mentir, en inventant une attaque contre un hôpital parisien. Face à ce gâchis financier et surtout humain, face à toute cette violence que vous n'avez pas su ou pas voulu maîtriser, parce que vous manquez de dignité républicaine, vous refusez de quitter la table. Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que vous devriez au moins présenter vos excuses aux policiers, aux « gilets jaunes » sincères et à l'ensemble des Français

Je vous remercie

pour le groupe Les Indépendants Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me félicite de la tenue de ce débat sur l'avenir de la politique agricole commune, quelques semaines avant les élections européennes. C'est en effet le moment opportun pour rappeler toute l'importance de l'agriculture et des agriculteurs en Europe et en France. La PAC est sans conteste une politique européenne stratégique, confrontée à de nombreux défis, qui devra être fermement défendue par les futurs députés européens français tout au long de leur mandat, et ce dès leur entrée en fonction. En effet, les débats qui se sont tenus au Parlement européen sur l'avenir de la PAC ont été mis en suspens avec le renouvellement des institutions et n'ont pas abouti à un vote en séance plénière. Seule la commission de l'agriculture a adopté sa position : elle est équilibrée et tente de mieux refléter les attentes des agriculteurs et des consommateurs, comme le fait d'ailleurs cette proposition de Du côté du Conseil, nous ne pouvons que constater des divisions profondes entre États membres. La France devra se montrer plus que jamais convaincante dans les prochains mois pour que ses partenaires la soutiennent, afin d'aller dans le sens du maintien d'une PAC commune et ambitieuse. Les cartes restent donc sur la table. Tout est encore possible pour l'avenir de notre agriculture européenne, le meilleur comme le pire, et les risques pesant sur l'avenir de la PAC demeurent omniprésents. La vigilance sera primordiale pour éviter tout détricotage de la politique agricole commune lors des négociations à venir entre le Parlement européen et le Conseil.

une variable d'ajustement du budget européen, alors qu'elle est le ciment de l'architecture européenne. Nous ne devons pas oublier que l'Europe est avant tout une puissance agricole : son budget ne doit pas être sacrifié sur l'autel des nouvelles priorités européennes par manque d'ambition budgétaire des États membres. Au contraire, nous devons davantage soutenir nos agriculteurs, qui font face à de nombreux défis : des normes de plus en plus exigeantes et de nouvelles demandes des consommateurs. L'alimentation de qualité est un enjeu majeur de nos territoires et sociétés. La concurrence est de plus en plus rude face aux autres puissances agricoles mondiales, les enjeux climatiques et environnementaux sont de plus en plus prégnants. Face à cette situation, il est primordial de préserver et protéger notre agriculture, mais aussi de la renforcer en la rendant plus compétitive, tout en préservant l'environnement. Il faut donc l'accompagner dans sa transition et son évolution, ce qui demande des moyens adéquats et des réponses adaptées. Nous l'avons déjà fait avec la loi Égalim ; il faut poursuivre ce travail et veiller à ce que les mesures adoptées soient bien mises en oeuvre sur toute la chaîne alimentaire. Il faut aussi que la future PAC accompagne la transition vers une meilleure répartition de la valeur entre le producteur, le transformateur et le distributeur. Il convient également d'adapter le droit de la concurrence aux spécificités agricoles de lutter davantage contre les pratiques déloyales de firmes internationales et transnationales. Il est également primordial de soutenir les petits agriculteurs, qui représentent le coeur de l'agriculture européenne, comme ceux qui se trouvent dans des zones à handicaps naturels. La Commission le propose déjà dans ses textes ; il faut aller plus loin, ainsi que sur les mesures valorisant les externalités positives de l'agriculture au regard des services qu'elle rend à la société et à l'environnement. l'installation des jeunes agriculteurs doit constituer un pan primordial de cette politique. Je me félicite d'ailleurs de la récente initiative prise par la BEI et la Commission pour lancer un programme européen visant à financer à hauteur de 1 milliard d'euros des prêts à taux réduits destinés aux jeunes agriculteurs. Cela contribuera au renouvellement indispensable des générations dans le monde agricole. Enfin, l'innovation doit être au coeur des priorités de l'agriculture de demain. Les moyens mis en place sont un signe positif de la volonté d'accompagner les agriculteurs dans cette transition. Il faudra que cela soit une opportunité pour eux et non pas un fardeau supplémentaire. Finalement, la nouvelle réforme de la PAC doit être considérée comme une occasion de nous poser la question du modèle agricole européen que nous souhaitons pour l'avenir : l'agriculture doit rester une priorité européenne, au vu de ses enjeux économiques, territoriaux et environnementaux. Nous devons réfléchir ensemble, avec nos partenaires, pour trouver les meilleures voies et les moyens budgétaires adéquats qui permettront de remplir ces objectifs. Dans le contexte du Brexit, une attention particulière devra aussi être portée à la préservation des relations commerciales futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, en veillant avant tout à préserver les intérêts des agriculteurs français et européens. Le groupe Les Indépendants soutiendra bien évidemment cette

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà maintenant près d'un an, le Sénat votait sa deuxième proposition de résolution européenne sur la réforme de la politique agricole commune. Nous étions alors nombreux sur ces travées à juger que le débat s'engageait sur des bases extrêmement inquiétantes. Aujourd'hui, force est de le constater, ces inquiétudes ne sont pas levées, tant s'en faut. La première d'entre elles porte évidemment sur les ressources budgétaires allouées à l'agriculture européenne. Le projet de de cadre financier pluriannuel de 2021 à 2027 marque à ce titre une véritable rupture, en prévoyant des coupes d'un niveau inégalé, bien supérieur aux 13 milliards d'euros correspondant correspondant au Brexit. C'est ainsi qu'une baisse de 15 % est proposée, ce qui représente un manque à gagner de près de 7 milliards d'euros pour l'ensemble de la ferme France et engage la pérennité des filières les plus fragiles, ainsi que la survie économique de nombre d'exploitations à travers notre pays. Le Gouvernement, sitôt ces annonces connues, s'est bien sûr empressé de contester ce déclin de l'ambition agricole de l'Europe. La vigueur de sa réaction ne saurait toutefois faire oublier à quel point elle fut tardive. En effet, focalisé sur le financement de nouvelles politiques européennes, le Gouvernement a relégué l'agriculture au second rang des priorités françaises durant les discussions budgétaires préparatoires. En refusant de jouer son rôle de premier défenseur de la PAC auquel nos partenaires étaient habitués, il a donné blanc-seing à la Commission pour proposer l'atrophie des crédits agricoles.

Cette erreur est lourde de conséquences, car chacun sait qu'une fois posées les bases d'une négociation il devient très difficile d'en inverser totalement les paradigmes. Tous les grands pays producteurs de la planète mènent une politique stratégique de renforcement de leurs concours publics à l'agriculture,

La question financière, pour centrale qu'elle soit, ne doit cependant pas nous conduire à ignorer l'autre sujet de préoccupation de cette réforme de la PAC, à savoir le nouveau modèle de mise en oeuvre proposé par la Commission elle-même au travers de l'élaboration par les États membres de plans stratégiques nationaux. Bien sûr, nous sommes tous en faveur d'une meilleure application du principe de subsidiarité, et nous savons tous que la PAC ne peut faire l'économie d'une simplification administrative supplémentaire. Toutefois, gardons à l'esprit qu'il doit s'agir avant tout de simplifier la vie des agriculteurs et non pas celle de la Commission, qui cherche surtout ici à se défaire d'une charge administrative en la transférant aux États membres. Absolument ! Le principal danger de cette proposition, qui couvre tant les actions du premier que du second pilier, est ailleurs : il réside en premier lieu dans la remise en cause de la gestion partagée de la politique agricole au niveau communautaire. Ne nous y trompons pas, ce qui en résultera précisément est bel et bien une renationalisation rampante de la PAC et la transformation de ce qui est aujourd'hui une politique commune cohérente en un simple supermarché de possibilités et d'outils. En effet, ce cadre global relâché, combiné aux nouvelles flexibilités accordées aux États membres, laisserait à chaque pays des marges de manoeuvre extrêmement importantes, qu'il s'agisse des règles d'éligibilité des bénéficiaires, des contrôles et des sanctions, du choix des types d'aides et de leurs montants, ou encore du niveau même de transferts financiers entre les piliers. Dans ce contexte, je ne peux que m'inquiéter du fait que cette nouvelle architecture à l'utilité plus que douteuse et au risque bien établi ne fasse pas l'objet d'une opposition plus résolue, notamment de la part des autorités françaises, qui me paraissent à ce sujet bien passives. Monsieur le ministre, c'est avec une gravité certaine que nous devons aborder la suite de ces négociations, dont vous avez hérité. C'est la légitimité même de la PAC et son efficacité au travers d'une mise en oeuvre cohérente sur l'ensemble du continent et le niveau de ses ressources budgétaires qui risquent d'être irrémédiablement remises en cause. La parole

une PAC impulsée par le Gouvernement, au service des agriculteurs et des biens communs européens. Cela exige notamment une contribution au développement des territoires fragiles dans l'Hexagone et outre-mer.

sénateurs, les maires, les conseillers départementaux et les députés européens ont cherché inlassablement à connaître le détail de la cartographie des zones soumises à contraintes naturelles et des zones soumises à contraintes spécifiques. En vain ! Puis cette carte est apparue au détour d'une réunion du Conseil national d'évaluation des normes, qui se tenait au Sénat. Est-ce normal ? Non, je ne le crois pas ! La carte en main, nous avons cherché à en connaître les données pédologiques pédologiques ou biophysiques et les critères sélectifs ayant permis d'y faire entrer un grand nombre de communes, mais aussi d'en sortir brutalement de nombreuses autres, comme c'est le cas dans mon département de l'Aude et dans celui du Gers. Las, ni vous, ni moi, ni même la Commission européenne, ne sommes en mesure d'obtenir les critères ayant permis à ce gouvernement de faire des choix aux conséquences vitales pour nos agriculteurs et nos communes. Quelles sont les données dont nous disposons aujourd'hui ? Pour les zones soumises à contraintes naturelles, c'est l'utilisation des données anciennes qui a prévalu. Pour l'exercice d'affinement économique qui aurait pu permettre de lisser la carte, vous avez choisi l'échelle des petites régions agricoles, échelle datant de 1946. Quelle logique ! Aujourd'hui, les PRA sont un ensemble économiquement hétérogène, notamment dans le Gers, et une cartographie basée sur de telles données est immanquablement discriminatoire. Je pourrais aussi vous parler du recours au recensement agricole et du calcul de la surface agricole utile, mais je ne dispose que de cinq minutes Pour les zones soumises à contraintes spécifiques, pour lesquelles vous disposiez d'une marge de manoeuvre plus large, le critère du maintien de l'activité touristique a été omis, ce qui est regrettable. Comme une résolution européenne du Sénat dont je suis l'autrice vous y invitait, vous pouviez utiliser le critère de continuité territoriale pour intégrer dans le zonage à contraintes spécifiques des territoires plus étendus, et non uniquement des communes isolées, territoires qui se trouvaient jusqu'ici exclus de la cartographie des zones défavorisées simples. Ce choix était à votre discrétion, mais vous ne l'avez pas retenu. Pourquoi ? Venons-en aux conséquences de telles décisions. Elles sont économiquement et socialement dramatiques, pour les agricultrices et les agriculteurs pour les exploitations les plus fragiles, dont bon nombre seront amenées à disparaître, ce qui amplifiera encore la désertification rurale. Monsieur le ministre, derrière un point sur la carte se dessinent de véritables drames humains. Quand cesserez-vous de les ignorer ? Que va-t-il advenir face à l'appauvrissement de ces territoires ? Je pense aux élus de la Piège, dans l'Aude, qui, à l'annonce de l'exclusion de leurs communes de la cartographie, ont placé, à l'entrée de leurs agglomérations, des écriteaux « Village à vendre ». L'incompréhension des éleveurs

Monsieur le ministre, où sont ces données ? Pourquoi refuser de les communiquer ? La justice administrative a été saisie. Le ministère a donné des informations, quand il a bien voulu donner les bonnes ! C'est insuffisant ! S'agit-il d'éviter les recours devant le tribunal administratif ? Vous l'avez dit, le Gouvernement a prévu d'accompagner les territoires et les agriculteurs qui sortiront du zonage à partir de 2019, sur une période de transition de deux ans, pour lisser les effets de la réforme. Et après, plus rien plus rien ? La sortie de la cartographie des zones défavorisées implique pour les producteurs agricoles la caducité des agréments sanitaires nécessaires pour la vente des produits issus de circuits courts au-delà d'une distance de 80 kilomètres. 80 kilomètres. Par ailleurs, la sortie du zonage entraînera de lourdes conséquences financières pour les jeunes agriculteurs, qui perdront alors la bonification de leur aide à l'installation. La question de l'ICHN, inhérente à la prise en compte des inégalités territoriales, dont l'hyper-ruralité souffre tout particulièrement, justifie une action résolue des pouvoirs publics français. Les difficultés que je viens de soulever

? Elle a permis, en l'espace de soixante petites années, de garantir une alimentation de qualité et en quantité suffisante pour tous les citoyens européens. N'en déplaise aujourd'hui aux vendeurs de peurs, ceux qui ont le ventre plein et la mémoire courte Comment réfléchir à l'avenir de l'Europe sans penser à une politique agricole qui façonne notre modèle de développement, aussi bien sur les plans stratégique, économique et environnemental, qui dessine notre modèle alimentaire, y compris dans sa dimension sanitaire, qui impacte l'aménagement de nos territoires ruraux et constitue, en définitive, une partie de notre identité ? Henri Cabanel disait qu'un agriculteur se suicide tous les deux jours. C'est un drame. L'émotion que cela devrait susciter est la même que celle que nous avons ressentie lorsque la charpente de Notre-Dame brûlait. C'est notre identité la plus profonde qui est touchée. Sans la PAC, permettez-moi d'affirmer qu'il n'y aurait sans doute pas l'Union européenne que nous connaissons. Pour la famille gaulliste qui est la mienne, la PAC est l'un des acquis couple franco-allemand voulu par Adenauer et de Gaulle. Ses difficultés actuelles sont le signe d'un affaiblissement de cet axe franco-allemand que le Président de la République s'était pourtant engagé à relancer. Tout l'enjeu des négociations en cours sur l'avenir de la PAC, sur la question tant du budget que de son contenu, est de définir quelle agriculture européenne, mais, plus généralement, quelle Europe nous voulons pour demain. Car, oui, monsieur le ministre, nous voulons l'Europe ! Ces négociations ont débuté en 2018 et ont suscité de vives inquiétudes dans nos campagnes. Au-delà du budget, préoccupation majeure plusieurs fois évoquée, le risque le plus important et le plus inédit est celui de la renationalisation de la PAC, qui fait craindre une course au moins-disant social et environnemental au détriment de nos agriculteurs, et qui est l'inverse de l'esprit européen. La situation est historiquement grave ; si nous en sommes là, monsieur le ministre, c'est que la négociation à laquelle a participé la France a été un échec. Le Président de la République a clairement sa part de responsabilité dans cet échec-

». Deux ans plus tard, nous y sommes. Les annonces présidentielles ont été mises en oeuvre. Et, comme l'a dit Jean Bizet il y a quelques instants, la direction prise sera difficile à modifier. Certes, entre-temps, plusieurs prises de paroles officielles, dont la vôtre, monsieur le ministre, ont dénoncé tant le budget que la réforme proposés pour la PAC. Le discours que vous nous avez tenu est volontariste, et je vous crois sincère. Mais je ne savais pas que nous étions en cohabitation, tant votre discours est différent de celui du Président Les négociations sont au point mort, nous dit-on. Et force est de constater que la France est étonnamment isolée au niveau européen. Le travail diplomatique de conviction et d'alliance doit être repris l'heure est venue d'obtenir des résultats. Ce n'est pas une question de majorité politique en Europe- vous le savez, monsieur le ministre. C'est une question de force et de présence de la France dans les instances de décision européennes. De ce point de vue, j'attire l'attention des électeurs du 26 mai prochain soyons vigilants s'agissant des groupes politiques européens auxquels les eurodéputés français vont adhérer ; car être dans l'opposition d'extrême ne sert à rien, sinon à affaiblir la position de la France. Ne pas dire où l'on siégera, et être ainsi nulle part, c'est très inquiétant. Les auteurs de la proposition de résolution se refusent à la fatalité d'un échec des négociations de la PAC. La procédure de décentralisation de cette politique doit être rejetée de manière unanime, au regard des risques qu'elle présente. Il faut défendre, à la place de cette procédure, un renforcement des mécanismes contracycliques et une meilleure mobilisation de la réserve européenne de crise, tant attendue par nos agriculteurs, afin de couvrir ces derniers contre les aléas économiques, climatiques ou géopolitiques. Il serait également juste et nécessaire de garantir une concurrence loyale et équilibrée protégeant nos produits alimentaires des importations.

de notre indépendance géostratégique et de notre sécurité alimentaire. Les négociations vont reprendre, après les élections européennes ; c'est un moment historique. Et je vous souhaite- je nous souhaite et je souhaite à la France -force, courage et réussite

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le rapport de l'ONU sur la biodiversité rendu public hier, et ce matin dans les journaux, donne à nos travaux de cet après-midi un éclairage tout à fait particulier. Un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, soit une espèce sur huit

Notre écosystème planétaire, condition non négociable de la survie de l'humanité, est à terme menacé si nous n'engageons pas un « changement profond » de nos modèles de production et de consommation. Nos modèles de production agricoles ne sont pas étrangers à ce dangereux déclin de la nature. Un seul exemple les engrais qui se déversent sur les côtes ont produit plus de 400 « zones mortes » dans les océans, ce qui correspond à une surface grande comme le Royaume-Uni. Dans un tel contexte, les grandes orientations de la future PAC apparaissent- pardonnez-moi l'expression -complètement à côté de la plaque. Nous ne pouvons pas nous satisfaire, pour cette grande politique intégrée de l'Union européenne, du simple replâtrage administratif qui nous est proposé. De ce point de vue, je ferai miens les mots de notre collègue eurodéputé Éric Andrieu : « La PAC a besoin d'une révolution et non d'un jusqu'en 2025. Cette révolution doit permettre de répondre aux grands enjeux qui sont face à nous : la protection de l'environnement, mais aussi le changement climatique, la santé humaine, la crise agricole actuelle. Les réponses à ces défis ne peuvent plus s'inscrire dans la continuité de celles apportées depuis 1992 ; autrement dit, elles ne sauraient continuer à favoriser une agriculture productiviste au service de l'agroindustrie. Nous payons tous, collectivement, les externalités négatives de ce système agroindustriel en payant pour la dépollution de l'air ou de l'eau, sans parler de la facture pour notre santé. Si le coût de la PAC représente 0,5 % du PIB européen, le coût des dépenses de santé s'élève à 10 Le lien entre alimentation et santé n'est plus à démontrer : pesticides, perturbateurs endocriniens, montée de l'obésité ... Cette révolution pourrait se matérialiser dans le nom même de la PAC, l'ajout d'un second « A », pour « alimentation ». Elle devrait se concrétiser à travers des aides publiques permettant une montée en gamme des productions agricoles et une transformation des modèles agricoles, cela afin de redonner un revenu décent aux paysans et de produire une alimentation plus saine, assortie d'un meilleur bilan carbone, dans des conditions respectant davantage l'environnement et le bien-être animal. Mais tout cela ne peut être fait sans une véritable ambition de la part de l'Union européenne. À cet égard, la baisse du budget de la PAC, qui va bien au-delà des effets mécaniques du Brexit, est plus qu'alarmante. Au commissaire à l'agriculture, Phil Hogan, qui demandait comment nous justifierions

La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui, qui rappelle les préconisations de nos deux précédentes résolutions, balaye bien le champ de ces différents enjeux et des réponses qu'il faut y apporter. C'est pourquoi notre groupe lui apporte son plein soutien. le Gouvernement entendra-t-il ce nouvel appel du Sénat à une autre ambition pour la politique agricole commune et renouera-t-il avec le volontarisme dont la France avait fait montre pour la soutenir dans les années précédentes ? La parole

L'agriculture est dans une passe difficile. Or ni l'Europe ni la France n'ont su répondre récemment à ces difficultés.

ce qu'espèrent un certain nombre de grandes puissances comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, qui voient bien sûr d'un mauvais oeil se construire cette Europe, qui avait su conduire une politique agricole commune.

; la France perdra sa place dans l'agriculture européenne. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, et nous avons besoin du Président de la République pour soutenir l'agriculture française.

les détracteurs de l'agriculture ne se rendent pas compte de ce que voudrait dire une pénurie de produits alimentaires. Sur le plan de la sécurité même de l'Europe et en particulier de la France, cette valeur stratégique

la vocation même de la politique agricole commune, qui était certes d'assurer une alimentation de qualité et à un prix correct pour l'ensemble des Européennes et des Européens, mais aussi de garantir un revenu aux agriculteurs,

parce qu'elle est essentielle pour assurer la souveraineté alimentaire de l'Europe, mais aussi parce que l'agriculture a un impact majeur sur l'environnement, qui est aujourd'hui un sujet d'urgence absolu. Le dernier rapport de l'IPBES nous l'a montré : la biodiversité, dont nous sommes dépendants pour notre existence même, est en grave danger. L'agriculture est bien un enjeu stratégique à cet égard : elle peut permettre la conservation, la préservation, voire le renforcement de la biodiversité, mais elle peut aussi, par l'usage des pesticides

pour revendiquer des moyens forts pour la PAC, il faut légitimer son budget et donc s'assurer qu'il répond aux attentes des citoyens en faveur d'une agriculture paysanne respectueuse de l'environnement. C'est pourquoi nous proposons d'inclure la notion de paiements pour services environnementaux

un outil pertinent pour assurer la transition agricole et rémunérer les agriculteurs pour les services qu'ils rendent à la société. Parce qu'ils permettent de réorienter les fonds de la politique agricole commune vers des pratiques vertueuses, ces instruments doivent être au coeur de la future PAC. Je sais que le Gouvernement, comme de nombreux acteurs agricoles, s'intéresse aujourd'hui à cet outil. Pour cette raison, il me semble qu'il faudrait aller au-delà du fonds Horizon Europe, destiné à financer des projets de recherche et d'innovation, et intégrer les PSE dans la PAC même, moyen le plus efficace pour garantir une rémunération mieux

de repli. Plutôt que d'appeler à ce que la rémunération des externalités positives de l'agriculture se fasse dans le cadre du fonds Horizon Europe, nous proposons de reprendre la rédaction adoptée par notre assemblée le 6 juin 2018 6 juin 2018 dans sa résolution européenne en faveur de la préservation d'une politique agricole commune forte, conjuguée au maintien de ses moyens budgétaires. Cet amendement a pour objet d'appeler à mieux rémunérer les services rendus par les agriculteurs à la société, mais sans lier cet appel au programme de développement et d'innovation qu'est le fonds Horizon Europe. Il est essentiel d'affirmer que la PAC doit avoir un rôle majeur dans la rémunération des services environnementaux plutôt que de rechercher les fonds dans d'autres budgets. Quel

le texte, n'est pas exclusive de la mise en oeuvre de PSE en dehors du cadre budgétaire de la politique agricole commune. commune. Compte tenu des baisses annoncées du budget de la politique agricole commune, il serait même plutôt préférable de financer les paiements pour services environnementaux

sur des thèmes parfaitement en phase avec l'objet d'éventuels PSE. J'ajoute- je ne l'ai pas dit ce matin en commission, mais je l'ai dit dans mon intervention en discussion générale - que le programme LIFE, qui est l'instrument financier de la Commission européenne pour tout ce qui concerne les projets relatifs à l'environnement et au climat, pourrait aussi contribuer au financement de PSE. La

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour renforcer les capacités de contrôle de l'application et de l'évaluation des lois, présentée par M. Franck Montaugé et plusieurs de ses collègues Dans la discussion générale, la parole est à M. Franck Montaugé, auteur de la proposition de résolution. Monsieur le président, monsieur

dans le prolongement des travaux que nous avions menés, en mars 2018, en présentant deux propositions de loi. La première d'entre elles était relative à l'amélioration des études d'impact des

Transmis à l'Assemblée nationale, ce texte n'a pas, à ce jour, été repris par elle. La seconde proposition de loi prévoyait la création d'un conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être, ainsi que la mise en oeuvre d'une démarche scientifiquement structurée d'évaluation des politiques publiques, ouverte à la participation effective des citoyens par des moyens appropriés. Jugée trop complexe, cette proposition de loi a été renvoyée voilà un an à la commission pour y être rediscutée. Elle ne l'a pas été, et nous avons souhaité, avec Jean-Pierre Sueur, Marc Daunis, Patrick Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, clore cette séquence de travail sur les fonctions du législateur par une proposition de modification du règlement de notre assemblée. Elle vise à nous permettre d'être plus plus efficaces dans le contrôle de l'application de la loi et l'évaluation de ses effets et, plus généralement, des politiques publiques, comme nous y enjoint l'article 24 de la Constitution de la V République. En effet, si le Parlement contrôle et évalue les politiques publiques de différentes manières, grâce notamment à l'instauration d'un espace réservé dans l'ordre du jour, à la possibilité de procéder à des contrôles « sur pièces et sur place de commissions d'enquête sur des sujets donnés et aux questions posées aux membres du Gouvernement, le contrôle de l'application des lois votées et promulguées peut être amélioré. Il est ainsi fréquent que les décrets et autres textes réglementaires nécessaires à l'application effective des lois soient publiés très tardivement ; parfois, ils ne le sont même ailleurs, de l'application sur le terrain, dans les territoires, de lois dont l'esprit initial, tel que voulu par le législateur, s'est transformé et a parfois été perdu en chemin, dans la chaîne administrative des interprétations ? Cet état de choses n'est pas acceptable, puisque la loi votée s'impose à toutes et à tous et qu'elle doit pouvoir s'appliquer dans des délais rapides dès lors qu'elle a été promulguée. Notre proposition de résolution initiale visait à compléter l'article 19 de notre règlement

d'un projet ou d'une proposition de loi. Sur le rapport de M. Philippe Bonnecarrère, dont je veux ici souligner la qualité du travail et la cordialité et que je remercie de m'avoir permis de participer aux auditions, la commission des lois a jugé que la création de ce droit de suite serait bienvenue, qu'il renforcerait utilement le suivi de l'application des lois, mais qu'il devait être assoupli. Sur ce point, les dispositions retenues par la commission des lois ne dénaturent pas la proposition de résolution initiale. Dès lors, si nous en décidons ainsi aujourd'hui, le rapporteur sera chargé de suivre l'application de la loi après sa promulgation et jusqu'au renouvellement du Sénat. Il pourra être confirmé dans ces fonctions à l'issue du renouvellement,

dans les mêmes conditions, un rapporteur pour assurer le suivi de l'application des dispositions relevant de leur domaine de compétence. Pour ce qui est de la mission d'évaluation des politiques publiques, notre position initiale n'a en revanche pas pu être conciliée avec celle de la commission. Nous proposions de faire figurer de manière explicite la notion d'« évaluation de la loi » dans notre règlement, dans le prolongement de la référence au « suivi de l'application de la loi ». La commission a jugé que le Parlement dispose d'une mission plus large d'évaluation des politiques publiques, qui relève déjà des commissions permanentes. C'est indéniable, mais qu'en fait-on en pratique ? Que l'évaluation des politiques publiques se distingue du suivi de l'application des lois, cela est certain. Reconnaissons qu'en toute logique on peut difficilement faire de l'évaluation sans en passer d'abord par un bilan de l'application des lois. La commission fonde aussi sa position sur le fait que l'évaluation est plus exigeante, qu'elle demande davantage de recul, qu'elle s'inscrit dans une démarche collective nécessitant la planification et la mobilisation de moyens spécifiques,

pour le moins songeur ... Différents groupes du Sénat, dont le mien et celui qui est conduit par le président Larcher, ont formulé, dans le cadre de la présentation du projet de révision constitutionnelle à la mi-2018, des propositions allant dans le sens d'une structuration de ce travail d'évaluation des politiques publiques. Je m'en réjouis. Parce que ce point est essentiel à mes yeux, je présenterai un amendement à l'article 1 visant à prendre en compte les remarques de la commission, pour que ne disparaisse pas purement et simplement de la proposition de modification de notre règlement l'évaluation des effets de la loi. Sans préjuger de l'organisation et des moyens internes au Sénat qui permettront d'y pourvoir, et en tenant compte -c'est un point important -des préconisations du Conseil d'État, rappelées en 2017 par son vice-président Jean-Marc Sauvé devant le groupe de travail de l'Assemblée nationale sur les moyens d'évaluation et de contrôle du Parlement, je proposerai que soit inséré à l'article 19 du règlement du Sénat les dispositions suivantes : « Dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, le rapporteur présente devant la commission une évaluation des premiers effets de la loi qui lui paraissent les plus significatifs. Dans les cinq ans après la promulgation de la loi, il doit être en mesure de présenter une évaluation complète de ses effets. Cette évaluation est effectuée au regard des motifs et de l'étude d'impact initiale de la loi. Elle prend en compte les effets de la loi sur les indicateurs de richesse légalement en vigueur et les objectifs de développement durable que la France met en oeuvre dans le cadre de ses engagements internationaux pour le climat et le développement. Elle indique les effets de la loi sur la trajectoire des finances publiques. Si nous adoptons cet amendement, nous ferons un petit pas de plus vers l'évaluation des politiques publiques. Dans le cas contraire, la question restera entière. J'ai bien conscience que le sujet est complexe et je constate qu'il suscite beaucoup de frilosité. Je crois cependant que le temps est venu,

que la conférence des présidents de chaque assemblée arrête un programme de contrôle et d'évaluation. Là aussi, notre assemblée a déjà réfléchi à cette question et formulé trois propositions : élargir à toutes

Monsieur le président, mes chers collègues, quel parlementaire n'est pas révulsé par les délais, d'apparence incompressibles, entre le vote des lois et leur application ? n'empêche d'ailleurs pas l'exécutif de se plaindre du temps perdu par les assemblées en débats et discussions d'amendements inutiles ! Faut-il, pour autant, en rendre responsables les sénateurs ou les députés, et leur donner une mission de « suivi »- de surveillance -de l'exécution des lois ? Je ne le pense pas.

du rapport, et non les parlementaires, dont la mission, n'en déplaise aux amateurs de procédures expéditives, est d'abord et toujours de faire la loi. Je crains en effet que, sur fond de réduction des effectifs et des moyens d'action des parlementaires, leur donner officiellement la responsabilité de contrôler la mise en oeuvre des lois qu'ils votent, loin de renforcer leurs pouvoirs, n'occulte encore un peu plus leur mission première : faire la loi. Le contrôle de l'action du Gouvernement, dont ils ont effectivement la charge, n'est pas le service juridique après-vente de la loi, mais l'évaluation de la manière dont celle-ci est exécutée sur le terrain. Le contrôle annuel, par la commission des lois, de l'état d'avancement de la production par l'exécutif des textes d'application des lois relevant de sa compétence me semble suffisant et correctement exécuté. Cela suffit à l'édification des citoyens, sans créer de surcharge pour la commission. J'ai une autre réticence, tenant au risque de spécialisation de quelques sénateurs de la majorité et de la minorité qui pensent comme elle. Par construction, un parlementaire est un généraliste ; la première vertu du Parlement, ce qui en fait autre chose qu'une assemblée d'experts, même juridiques, est qu'en théorie du moins la loi est le produit du débat collectif, et non d'échanges entre et non d'échanges entre spécialistes. Le fait que les non-spécialistes, ceux qui ne trouvent pas évidentes les certitudes d'habitude,

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues,

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, bien que son examen vienne s'inscrire un peu maladroitement dans l'ordre du jour, en anticipant les réformes du règlement proposées par le président du Sénat et les débats institutionnels à venir, ce texte de nos collègues du groupe constitue une proposition intéressante, destinée à renforcer le contrôle de l'application des lois. Il s'agit sans conteste de l'un des moyens à privilégier pour adapter l'action parlementaire aux contraintes institutionnelles qui s'imposent à nous, plus de soixante ans après la création de la V République. Il nous incombe, en effet, de trouver de nouvelles formes de réponses aux attentes de nos concitoyens à notre égard. Au-delà du regret d'une époque qui a vu naître le groupe du RDSE, nous sommes nombreux à considérer que le parlementarisme rationalisé n'a pas tenu toutes ses promesses. Certes, dans un premier temps, la clarification des bornes de l'action parlementaire a pu être jugée efficace. Avant cela, en effet, la pratique des décrets-lois avait fait couler beaucoup d'encre, tant dans les universités que place du Palais-Royal, jusqu'à l'avis du Conseil d'État du 6 février 1953, sur lequel s'est fondé le Constituant de 1958 pour rédiger l'article 34 de la Constitution. Cette évolution a permis de doter nos gouvernements d'une légitimité législative déterminante pour inscrire leur action dans la durée. Cependant, associé à un raccourcissement des échéances électorales, notamment au passage du septennat au quinquennat, mouvement contre lequel nous nous sommes élevés par le passé et restons mobilisés, ce nouvel équilibre institutionnel n'a pas permis d'éviter la dégradation de la qualité législative. La grande sophistication des règles d'irrecevabilité rend de plus en plus difficile l'examen des textes déposés par des parlementaires, ceux-ci devant se conformer à des considérations simultanées de budget, de calendrier et de fond auxquelles échappent les gouvernements. Je pense en l'espèce au respect du domaine réglementaire, dont les contours varient d'un code à l'autre ! Fondé sur les mêmes conclusions, le rééquilibrage institutionnel opéré par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 visait à renforcer la mission de contrôle du Parlement, en partant du principe que l'équilibre des pouvoirs nécessite que, quand l'initiative législative des chambres parlementaires est réduite au profit de l'initiative gouvernementale, celles-ci soient dotées de prérogatives de contrôle renforcées. Cela rejoint l'injonction du philosophe Alain : « Nous n'avons point à louer ni à honorer nos chefs, nous avons à leur obéir à l'heure de l'obéissance, et à les contrôler à l'heure du contrôle. Encore faut-il, mes chers collègues, que des heures soient effectivement dévolues au contrôle dans l'agenda parlementaire ... La révision de 2008 visait à aménager ces temps de contrôle, en en reconnaissant tout d'abord la valeur constitutionnelle, par la consécration de cette mission à l'article 24 de notre texte fondateur, à côté de la mission législative, et en adaptant l'ordre du jour en conséquence. Cependant, de nombreuses propositions du comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions piloté par Édouard Balladur sont restées lettre morte. Si tout le monde s'accorde sur la nécessité de renforcer le contrôle d'application des lois, il n'est point aisé de définir la forme adéquate. C'est ainsi que la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois a été supprimée trois ans seulement après sa création en 2011. La proposition de modification du règlement du Sénat qui nous est soumise aujourd'hui se rapproche toutefois davantage de l'esprit du Constituant. En effet, le comité Balladur de 2007 avait proposé d'« instituer dans les commissions permanentes des " équipes " de contrôle de l'exécution des lois, composées d'un parlementaire de la majorité et d'un parlementaire de l'opposition ». La solution retenue par le groupe socialiste et républicain vise à fractionner cette mission en la confiant, pour chaque texte, au rapporteur de celui-ci, au-delà de son adoption. Cette proposition nous paraît pertinente et nous y sommes favorables. Concernant l'évaluation de la loi, M. Bonnecarrère, dont je tiens à saluer le travail, minutieux et précis comme à l'habitude, propose d'ajourner l'examen de la question du renforcement de l'évaluation, afin de pouvoir parvenir à une solution plus étoffée : nous sommes convient d'insister sur le fait que cette modification n'apportera pas de réponses aux difficultés les plus sérieuses. Je citerai, à titre d'exemples, la faiblesse des études d'impact, qui ne nous permettent pas de procéder à une bonne évaluation, ou l'absence de voies d'action en justice en cas de constatation d'une mauvaise application

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis le début des années soixante-dix, le Sénat procède au contrôle de l'application des lois. Comme le soulignait le président Gérard Larcher dans sa conférence de presse du 24 janvier 2018, « le retard pris dans l'application des lois est un des principaux dysfonctionnements de notre République

avec les autres travaux : l'exercice du droit de suite du rapporteur aurait vocation à alimenter le bilan annuel de l'application des lois, non à s'y substituer. En outre, les commissions permanentes pourraient désigner plusieurs rapporteurs pour suivre l'application d'une loi. Enfin, le droit de suite ne concernerait pas les rapporteurs des commissions spéciales.

En outre, l'évaluation des politiques publiques se distingue du suivi de l'application des lois. Plus exigeante, l'évaluation demande également davantage de recul. Enfin, l'évaluation des politiques publiques s'inscrit dans une démarche collective, nécessitant la planification et la mobilisation de moyens spécifiques. Si le rapporteur du projet ou de la proposition de loi peut y participer, il peut difficilement en être le seul acteur. Mes chers collègues, il apparaît particulièrement important de renforcer le suivi de l'application des lois sans engorger les commissions permanentes. De même, il est pertinent de circonscrire le champ de ce texte au seul suivi de l'application des lois. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, de l'article 21 de la Constitution, « le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Dans la circulaire du 29 février 2008 relative à l'application des lois, constatant que « l'objectif consistant à prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires dans un délai de six mois suivant la publication de la loi [n'était] pas encore atteint », le Gouvernement rappelait l'obligation de résultat qu'il s'était fixé Selon le credo même du Gouvernement, « chaque disposition législative qui demeure inappliquée est une marque d'irrespect envers la représentation nationale et de négligence vis-à-vis de nos concitoyens ». Il résulte de l'inexécution des lois par le Gouvernement, en raison même de l'obligation à caractère constitutionnel qui s'impose à lui, que la responsabilité pour faute de l'État peut être engagée en cas de retard ou de carence dans l'application des lois. Qu'en est-il dans les Nous ne connaissons que trop cette réalité : il n'est pas rare que les décrets et autres textes réglementaires nécessaires à l'application effective des lois soient publiés très tardivement. lorsque le Parlement a autorisé les policiers municipaux à consulter directement le fichier des plaques d'immatriculation ou celui des permis de conduire, il a fallu plus de deux ans pour prendre le décret d'application. Hormis quelques expérimentations, la consultation de ces fichiers est toujours impossible, faute de moyens matériels. de moyens matériels. On en arrive à des situations absolument surréalistes, où l'expérimentation de la mise en oeuvre d'un décret d'application de portée générale intervient plus de deux ans après le vote de la loi On observe par ailleurs un certain nombre de carences dans l'application des lois. Maryse Deguergue, professeur de droit public à l'université ce titre que, dans certains cas, « ce n'est plus à proprement parler un retard qui est reproché au Gouvernement, mais une abstention qui équivaut, selon les termes mêmes des arrêts les plus récents, à un refus de satisfaire à l'obligation qui lui incombe De telles situations sont problématiques, car la loi votée doit pouvoir s'appliquer dans des délais rapides et s'imposer à toutes et à tous dès lors qu'elle a été promulguée. Rappelons une évidence : ces lois, dont l'exécution peine à être mise en oeuvre,

Disons-le franchement, comment le Gouvernement peut-il attendre autant des collectivités territoriales et prétendre au crédit de sa parole, s'il ne s'astreint pas à respecter l'obligation constitutionnelle d'assurer l'exécution des lois qui lui incombe ?

Au cours de l'histoire de notre République, le Sénat s'est présenté comme le pionnier du contrôle de l'application des lois. Cela fait ainsi plus de quarante ans que la chambre haute dresse un bilan annuel de l'application des lois, proposant une vision globale des efforts mis en oeuvre par le Gouvernement. Au printemps, chaque président de commission réalise un bilan de l'application des lois relevant des compétences de sa commission. Le président de la délégation du bureau du Sénat chargée du travail parlementaire, de la législation en commission, des votes et du contrôle élabore ensuite le bilan annuel de l'application des lois, publié à la fin du mois Enfin, le groupe de travail du Sénat sur la révision constitutionnelle propose de renforcer le suivi de l'application des lois, notamment en autorisant les présidents des deux assemblées, soixante députés ou soixante sénateurs à saisir le Conseil d'État en cas de retard ou de carence du Gouvernement. résolution que nous examinons aujourd'hui prévoit la création d'un droit de suite au bénéfice du rapporteur d'un texte, confiant ainsi à ce dernier la responsabilité de suivre l'application de la loi après sa promulgation et jusqu'au renouvellement du Sénat. Il est également prévu que les commissions permanentes puissent désigner, dans les mêmes conditions, un autre rapporteur à cette fin. Le rapporteur resterait libre d'organiser ces travaux de suivi, notamment en fonction du nombre de décrets manquants. Ses observations auraient vocation à alimenter le bilan annuel de l'application des lois, dont l'existence serait reconnue par le règlement du Sénat. Les travaux de la commission des lois ont par ailleurs permis d'expliciter la procédure applicable aux textes examinés par une commission spéciale. Les commissions permanentes seraient ainsi habilitées à désigner un rapporteur pour suivre l'application des dispositions relevant de leur domaine de compétence. Je salue les travaux menés par la commission des lois, en particulier par notre collègue Philippe Bonnecarrère,

En effet, s'il apparaît que la création d'un droit de suite au bénéfice du rapporteur est susceptible de renforcer utilement le suivi de l'application des lois, il est aussi de notre devoir de veiller à ce que cela ne conduise pas à engorger les commissions permanentes.

L'article 24 de la Constitution dispose, depuis 2008, que le Parlement « évalue les politiques publiques ». Or l'évaluation de la loi n'est pas exactement la même chose : le Parlement fait la loi, tandis que le Conseil constitutionnel en évalue la constitutionnalité. Dans une décision du 2 janvier 2002 relative à la saisine de la loi de modernisation sociale, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs réaffirmé la nécessité, pour le législateur, Les implications des dispositions de l'article 24 sont donc substantiellement différentes de celles qui ressortent de la formulation de la proposition de résolution. Les amendements permettent de remédier à cette difficulté conceptuelle en recentrant la proposition de résolution sur le suivi de l'application des textes plutôt que sur leur évaluation

C'est pour cette raison que je partage l'idée du vice-président Jean-Pierre Sueur de rendre obligatoire l'inscription dans l'année à l'ordre du jour des propositions de loi adoptées par l'autre assemblée. En tout état de cause, le Sénat agit déjà, à travers les commissions permanentes, pour assurer un suivi de l'application des textes législatifs examinés en commission. Ce travail est indispensable dans la mesure où le Parlement est tributaire de l'exécutif, les textes d'application définissant dans la plupart des cas la mise en oeuvre des lois.

Je crois qu'en la matière il serait utile de réfléchir à des dispositifs qui permettent au législateur de mieux contrôler l'application de la loi par l'exécutif. Bien sûr, à titre individuel, les parlementaires peuvent solliciter le ministre concerné ou poser une question orale ; à titre collectif, ils peuvent mettre en place des mécanismes de contrôle de l'application et d'évaluation, par le biais de rapports ou de missions temporaires. Cela me paraît néanmoins insuffisant au regard de l'enjeu démocratique. Il est impératif qu'un texte de loi soit strictement conforme à ce qui a été décidé par la représentation nationale. Pourquoi ne pas envisager la possibilité d'une saisine parlementaire exceptionnelle dans le cas où un décret d'application n'est pas conforme au texte

Pour le reste, je me joins aux propositions du groupe de travail du Sénat sur la révision constitutionnelle, en particulier en ce qui concerne le renforcement des capacités d'évaluation des commissions permanentes.